contre. Acte est donné de votre mise au point. Elle sera publiée au et figurera dans l'analyse politique du scrutin concerné. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi de programmation, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des affaires étrangères, messieurs les rapporteurs, monsieur le rapporteur pour avis, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, il y a quelques semaines, j'ai participé à Berlin à une rencontre de la Coalition pour le Sahel. Il y a quelques jours, je me suis rendu en Inde, où j'ai eu des échanges nourris au sujet de la COP26 sur le climat, qui se tiendra l'automne prochain à Glasgow. Mardi et mercredi derniers, je me trouvais à Londres, pour une réunion du G7. Autant de rendez-vous internationaux qui m'ont permis de constater que le nouvel élan que nous sommes en train de donner à notre politique de développement solidaire, grâce au projet de loi qui nous rassemble aujourd'hui, est un nouvel élan pour l'ensemble de notre diplomatie. La réponse à chacune des questions essentielles que j'ai abordées avec mes interlocuteurs de Berlin, de Delhi et de Londres passe, en effet, par le développement de la solidarité internationale. C'est la clé pour rendre des perspectives d'avenir aux populations du Sahel après plus de huit années d'instabilité et de violence. C'est la clé pour tenir les objectifs de l'accord de Paris et renforcer la résilience des pays les plus exposés aux premiers effets des dérèglements climatiques. C'est la clé d'une relance durable, pour tirer tous les enseignements de la crise pandémique. C'est pourquoi le texte que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui consacre notre politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales comme un pilier à part entière de notre politique étrangère. C'est pourquoi il renforce et perfectionne les leviers d'action qui nous sont devenus indispensables pour faire face à la nouvelle donne internationale. C'est pourquoi il constitue une étape décisive dans la refondation, au service des Françaises et des Français, d'une diplomatie des résultats, d'une diplomatie du XXI siècle, d'une diplomatie des valeurs. Une diplomatie des résultats, car, dans un monde d'interdépendances, la solidarité internationale est un impératif d'efficacité en même temps qu'une question de justice. Aider les autres, c'est nous aider nous-mêmes. Je crois que chacun l'a bien compris depuis qu'une pandémie mondiale est brutalement entrée dans nos vies.

Depuis un an, j'y insiste. Nous avons constamment été à l'initiative avec nos partenaires européens et avec l'Organisation mondiale de la santé Plus de 50 millions de doses de vaccins ont ainsi déjà été distribuées Covax dans 121 pays, dont 72 pays en développement. La France joue un rôle capital au sein d'ACT-A pour, d'une part, promouvoir les transferts de technologie et les partenariats industriels, et, d'autre part, distribuer des dons de doses de vaccins, comme elle a commencé à le faire à titre national en Mauritanie. Il s'agit aussi pour la France de traiter de façon concrète et opérationnelle tous les goulots d'étranglement, singulièrement ceux de production, pour garantir la disponibilité des vaccins. Cela intègre, évidemment, les restrictions aux exportations ainsi que la levée des brevets. La France n'a pas de tabou à ce sujet, mais il ne s'agit pas d'en faire « la recette miracle comme cela a été trop rapidement et de façon parfois un peu simpliste mis en avant. L'urgence est bien la production. Les évolutions portées par ce projet de loi nous sont aussi nécessaires pour bâtir une vraie diplomatie du XXI siècle, ce siècle de défis communs. Face au covid, face à l'urgence climatique, face aux migrations, tous les pays, toutes les sociétés civiles ont un rôle à jouer. C'est dire que les solutions se trouvent aussi au Sud et que notre responsabilité est de veiller à ce qu'elles puissent y voir le jour. Oui, il y va de notre responsabilité, car ces défis engagent l'avenir : l'avenir de notre pays, l'avenir des nouvelles générations, l'avenir de la planète que nous avons en partage. Le développement solidaire, c'est enfin un instrument privilégié de la diplomatie des valeurs valeurs que nous voulons et devons mener aujourd'hui. Car certains, vous le savez, sous couvert de solidarité, cherchent en réalité à imposer à nos partenaires les plus vulnérables des conditions et des contreparties qui ne sont pas compatibles avec les exigences de souveraineté et de respect des droits fondamentaux que nous portons pour nous-mêmes, mais aussi sur la scène internationale. Notre intérêt- je le dis très clairement -n'est pas de voir ces exigences perdre du terrain dans la compétition des modèles lancée par les puissances autoritaires. Au contraire, notre intérêt est que ces exigences soient partagées par d'autres, à commencer par ceux des pays qui sont prioritaires dans notre aide publique au développement (APD). C'est aussi le sens de ce texte. À la différence de la précédente loi sur le développement, celle de 2014, le présent texte fixe une trajectoire budgétaire. Cette trajectoire nous permettra de concrétiser l'engagement du Président de la République de consacrer 0,55 % de la richesse nationale à notre aide publique au développement d'ici à 2022. Pour toutes les raisons que je viens de rappeler, nous avons fait le choix de garder le cap que nous nous étions fixé, en dépit des perturbations, notamment économiques, que nous traversons aujourd'hui, et ce contrairement à certains de nos voisins qui ont pris le chemin inverse. Je suis fier de ce choix, qui montre que nous continuons à nous projeter dans le temps long, qui est le temps du développement et des changements en profondeur dont nos partenaires ont besoin. Paradoxalement, les urgences de la crise actuelle sont d'ailleurs venues, à leur façon, nous rappeler la nécessité d'une transformation inscrite dans la durée. Il s'agit également d'un projet de loi d'ambition puisque son examen en première lecture à l'Assemblée nationale a permis de compléter l'article 1, en prévoyant que la France s'efforcera, en 2025, de consacrer à l'aide publique au développement 0,7 % de son revenu national brut, soit la cible fixée par les Nations unies.

de ce que signifie ce premier pas. Après le vote de l'amendement auquel je fais référence, sur le taux de 0,7 %, les organisations de la société civile ont salué un moment historique. De cela aussi, je suis très fier, d'autant plus fier que ce combat, comme vous le savez, n'était pas gagné d'avance. Ces moyens renforcés doivent permettre de faire une vraie différence sur le terrain.

afin d'obtenir des résultats tangibles que la représentation nationale pourra apprécier sur des bases objectives et détaillées, grâce à la création d'une commission d'évaluation indépendante rattachée à la Cour des comptes. Cette commission sera chargée de mesurer l'impact concret des projets que nous soutenons et de se prononcer sur l'efficacité de notre aide publique au développement. Puisque des moyens accrus vont être consacrés au développement, il est légitime que nos concitoyens sachent à quoi ils serviront. Je crois que nous serons tous d'accord sur ce point et je sais que nous partageons ce même objectif. Faire mieux, c'est d'abord clarifier nos priorités géographiques. Dans la continuité des décisions prises lors du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, le Cicid, en 2018, nous proposons d'orienter notre aide en dons sur 19 pays prioritaires qui concentrent les fragilités : Haïti et 18 pays d'Afrique subsaharienne.

qui articule engagement militaire, aux côtés des forces du G5 et de nos partenaires européens et internationaux, et soutien aux populations, sur tout l'arc de la solidarité internationale, qui va de l'humanitaire au développement, sans oublier l'étape cruciale de la stabilisation. Depuis quelques années, les moyens affectés aux pays du Sahel sont en constante augmentation. Entre 2016 et 2019, notre aide publique au développement en faveur des pays du G5 Sahel est passée de 382 millions d'euros à plus de 503 millions d'euros.

maintenu 200 000 enfants nigériens à l'école primaire et réhabilité près de 2 000 classes au Mali. Prises ensemble, ces avancées nous permettent de faire reculer durablement la menace terroriste au Sahel, qui est aussi- nous en sommes tous conscients -une menace pour la sécurité des Français et des Européens. Faire mieux, c'est aussi clarifier nos priorités thématiques autour de nos biens communs- la santé, mais aussi le climat et la biodiversité -, autour de ces formidables leviers de développement que sont l'éducation et l'égalité entre les femmes et les hommes, et autour d'un objectif global de lutte contre les fragilités, qui sont des facteurs d'instabilité pour les sociétés, et donc des facteurs d'instabilité pour le monde entier. Évidemment, ces sujets sont liés les uns aux autres. Faire mieux, c'est donc également veiller à les traiter comme un tout, pour répondre à la complexité des problèmes qui se posent sur le terrain et décupler l'efficacité de nos actions. D'où l'attention que nous apportons à des questions comme celles de la scolarisation des filles ou encore des interactions entre santé humaine et santé animale, qui sont au confluent de nos différentes priorités. D'où, pour ne prendre qu'un seul exemple, le soutien que nous apportons à la relance du projet de la « grande muraille verte » au Sahel, qui crée une dynamique vertueuse entre écologie et emploi des populations. Faire plus, faire mieux, mais aussi faire avec : avec nos partenaires du Sud, et pas simplement pour eux. C'est aussi cela, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, une diplomatie du XXI siècle. C'est pourquoi nous proposons également un changement de méthode. Nous voulons travailler autrement avec les pays du Sud, en particulier avec leurs sociétés civiles, pour bâtir et réaliser ensemble les projets dont les populations ont besoin. Nous voulons mieux valoriser le rôle des ONG françaises, auxquelles nous proposons de reconnaître un droit d'initiative. Nous voulons encourager la coopération décentralisée, qui permet à nos communes, à nos départements et à nos régions de partager leur expertise et leur expérience avec les collectivités locales des pays en développement. Nous voulons réinventer le volontariat de solidarité internationale en ouvrant ce dispositif emblématique à la jeunesse du Sud, qui pourra venir prêter main-forte à nos associations, ici, en France. Nous voulons mettre à contribution les diasporas africaines en France, qui sont des relais précieux entre la France et le continent africain. Dire que le développement est un pilier de notre politique étrangère a des conséquences très concrètes. Cela signifie que le pilotage par l'État de notre action dans ce domaine doit être renforcé et que cette action doit répondre à des impératifs stratégiques.

Ce texte prévoit ainsi la mise en place d'une chaîne de commandement et de responsabilité nettement réaffirmée, du plus haut niveau, avec le Conseil présidentiel du développement, qui s'est réuni pour la première fois en décembre dernier, jusque dans nos pays partenaires, où le rôle dévolu aux ambassadrices et ambassadeurs sera renforcé, dans le cadre d'un conseil local du développement qui rassemblera régulièrement, sous leur présidence, toutes celles et tous ceux qui contribuent à cette politique au quotidien, en lien direct avec les populations bénéficiaires. de passer, bien sûr, par nos opérateurs, notamment par Expertise France que nous voulons enfin intégrer dans le groupe AFD en vue de réarmer notre pays sur le terrain de la coopération technique, en l'articulant mieux avec la gamme de tous nos outils financiers : dons, prêts, garanties, etc. Nous pourrons ainsi agir avec toute la palette de nos instruments. Monsieur le président Cambon, pour répondre à votre préoccupation majeure, qu'avec l'ensemble de ces changements il s'agit, en un mot, de remettre le développement sur ses pieds, car- disons-le -notre politique de développement n'en est pas vraiment une tant qu'elle semble menée par les instruments qu'il lui revient d'utiliser. Je dois remercier le Sénat, qui a toujours fait preuve d'une grande vigilance sur ce point, notamment lors de l'examen des projets de loi de finances, afin qu'il n'y ait pas de confusion entre les objectifs politiques que nous visons et les moyens que nous mettons ensuite à disposition pour les atteindre. Cette Cette politique de développement solidaire, nous devons, dans la compétition des modèles qui fait rage aujourd'hui, la mettre au service d'une géopolitique des valeurs. Ce tournant, je le revendique : je pense, en effet, que nous n'avons rien à gagner à laisser le champ libre à ceux qui confondent délibérément aide au développement et mise au pas des sociétés. plus laisser le champ libre à ceux qui font du clientélisme vaccinal un levier de puissance. Si nous ne mettions pas à profit nos instruments de solidarité internationale pour proposer à nos partenaires du Sud une autre voie que celle de la dépendance, voire de la sujétion, nous commettrions une faute et une erreur. Ce serait une véritable faute et un manquement aux valeurs que nous portons de les laisser pris au piège d'un tête-à-tête avec des puissances prédatrices prêtes à bafouer leur souveraineté. Ce serait une très grave erreur- une erreur stratégique -de ne pas défendre, là où elles sont attaquées, les valeurs universelles qui font de l'horizon du développement durable, tel qu'il a été défini dans l'Agenda 2030 adopté par les Nations unies en 2015, un véritable horizon de progrès. Un horizon qui, indissociablement, lie ensemble la lutte contre la pauvreté, le combat pour la planète, la mise en commun des savoirs et de la recherche scientifiques, les libertés fondamentales et les principes de l'État de droit et de la gouvernance démocratique. À ce propos, je tiens à saluer l'amendement adopté sur l'initiative de l'Assemblée nationale qui permettra la création d'un dispositif de restitution des produits de cession des « biens mal acquis » et qui reprend une proposition de loi de de loi de Jean-Pierre Sueur, dont je salue le travail sur ce sujet. C'est un moyen très concret de lutter contre les ravages de la corruption et de la prévarication, qui s'inscrit parfaitement dans l'esprit de notre texte. Des précisions ont été apportées au cours de vos débats en commission ; je me félicite de ce travail constructif : il a permis de renforcer l'association des organisations de la société civile aux projets de développement financés par ce biais afin qu'ils bénéficient bel et bien aux populations concernées. Aujourd'hui, nous en avons de tristes exemples chaque semaine, cet horizon humaniste, qui est l'essence même du développement, est remis en cause par de nouveaux acteurs sans scrupules, notamment en Afrique. C'est l'un des aspects de la brutalisation de la vie internationale. Face à cet état de fait, notre intérêt- là aussi, de long terme -est de mobiliser les leviers de notre politique de développement solidaire, aux côtés de nos leviers d'action multilatéraux, pour faire vivre concrètement les valeurs que nous voulons voir au centre du monde de demain. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que davantage d'organisations internationales s'implantent en France. Ce projet de loi vise donc aussi à renforcer l'attractivité de notre pays, notamment en simplifiant et en accélérant l'octroi des privilèges et immunités, pour renforcer notre capacité d'influence. Ces deux mouvements sont complémentaires. Madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, vous m'avez entendu y faire allusion à plusieurs reprises, le texte qui vous est soumis aujourd'hui s'est enrichi au fil des échanges que j'ai eus, en février, avec vos collègues de l'Assemblée nationale. Vous-mêmes, vous vous en êtes pleinement saisis dans le cadre de vos travaux en commission des affaires étrangères, mais également, monsieur Requier, en commission des finances.

Dans ce travail collectif, qui s'inscrivait dans le prolongement de plusieurs années de réflexion et de discussions extrêmement fructueuses menées avec la représentation nationale, sous l'égide de la regrettée Marielle de Sarnez et du président Cambon, et les organisations de la société civile, de la société civile, j'ai vu un très beau signal, confirmé par le vote du texte à l'unanimité en première lecture à l'Assemblée nationale. Un signal à l'adresse de nos partenaires du Sud et de la communauté du développement, bien sûr, mais aussi, et même avant tout, un signal à l'égard des Françaises et des Français. À mes yeux, le consensus qu'ils ont vu se dessiner fait honneur à notre démocratie. Il répond, de manière pragmatique, à la nécessité de regarder en face les bouleversements du monde, pour leur apporter des solutions efficaces avant qu'ils ne viennent percuter notre quotidien, comme l'a fait la crise pandémique. Dans un monde également bouleversé, trop souvent, par une forme de perte de sens, il répond à notre volonté, que vous partagez- j'en suis certain -, de redonner un sens concret aux valeurs qui nous sont chères : la solidarité, le progrès, une certaine idée de l'humain et de sa dignité. mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, que vous aurez à coeur de travailler avec moi à renouveler, en le faisant vôtre, ce signal de responsabilité et de détermination. La parole

mes chers collègues, c'est aujourd'hui une satisfaction de pouvoir débattre de ce projet de loi relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, que nous attendions depuis plus de deux années. Notre commission suit depuis longtemps cette politique avec beaucoup d'attention, car les enjeux en sont essentiels. En particulier, ni la France ni l'Europe ne peuvent se désintéresser de la situation du continent africain, notre voisin. Le texte transmis au Sénat comporte, monsieur le ministre, de nombreuses avancées. Notre commission s'est toutefois efforcée de l'améliorer sur plusieurs points. D'abord, ce projet de loi dit « de programmation » ne couvre en réalité que l'année 2022. Cela nous a paru insatisfaisant et nous nous sommes efforcés d'y remédier. Certes, les incertitudes de la situation économique rendent l'exercice délicat. Nous sommes partis des prévisions du FMI (Fonds monétaire international), pour dessiner une trajectoire avec des marches annuelles d'environ 800 millions d'euros. Parallèlement, nous avons prévu un rendez-vous en 2023, pour réviser cette évolution en fonction de la conjoncture et, éventuellement, remettre au premier plan les 0,7 % du RNB Nous pourrons toutefois débattre de la forme exacte de cette programmation, notamment à l'occasion d'un amendement qui sera présenté par le rapporteur pour avis de la commission des finances. Par ailleurs, le volume de nos engagements financiers ne doit pas constituer l'alpha et l'oméga de cette politique de développement solidaire. Le choix des pays vers lesquels nous orientons nos financements, la nature des projets financés, la manière même dont nous les finançons sont tout aussi importants. Ainsi, seulement 18 % de notre aide dite « pays programmable » va vers les pays les moins avancés, quand la plupart de nos partenaires sont à 30 % ou à 40 %.

Notre commission a adopté des amendements pour remédier à cette situation de manière progressive. Ils permettront de recentrer notre aide au développement sur les pays qui en ont le plus besoin ainsi que sur les services essentiels : éducation, santé, agriculture et alimentation. Car notre aide au développement s'est parfois un peu égarée en s'efforçant de maximiser les volumes de prêts, le plus souvent à taux de marché, au bénéfice des pays émergents. Si les apports de notre commission peuvent conduire à stabiliser, voire à freiner un peu l'activité bancaire de l'AFD (Agence française de développement) au profit de sa gestion des dons, nous l'assumons. Il s'agit aussi de redonner du sens à cette politique et de la rendre plus lisible pour nos concitoyens. Troisième sujet, traité selon nous de manière incomplète par le projet de loi : la question du pilotage et de la gouvernance de cette politique. des comptes, dans son rapport de 2020 sur les opérateurs de l'action extérieure de l'État, en a souligné la complexité actuelle. Les instances de direction, de concertation et de consultation sont nombreuses, leurs missions enchevêtrées. Les dispositions qui figurent au sein du cadre de partenariat global annexé n'apportent pas de simplification majeure dans ce domaine. Notre commission a donc adopté des modifications afin de réaffirmer le rôle prééminent du ministre chargé du développement. Nous saluons cependant la création d'un conseil local du développement, placé auprès de l'ambassadeur. Il contribuera à l'un des impératifs que nous souhaitons particulièrement souligner : celui d'un meilleur alignement de notre politique de développement solidaire, non seulement avec les orientations de la diplomatie française, mais aussi avec nos autres politiques publiques. Car l'aide au développement ne doit pas être coupée de nos propres réalités. L'« Équipe France » doit promouvoir de manière cohérente nos objectifs de solidarité avec ceux qui sont les nôtres en matière de développement économique, de sécurité globale ou encore de rayonnement de la langue française au travers du soutien à son apprentissage. Autre apport majeur du texte, la création d'une commission indépendante d'évaluation de la politique de développement solidaire. Il s'agit là d'une de nos préconisations de longue date. Le nouvel organisme, inspiré de la commission d'évaluation britannique, possédera à la fois l'indépendance et l'expertise technique. Il fournira ainsi au Gouvernement, mais aussi au Parlement, les éléments pour instaurer un véritable « pilotage par les résultats ». Nous avons souhaité mieux définir la composition de ce nouvel organisme, en entérinant son placement auprès de la Cour des comptes, gage d'indépendance, mais aussi en prévoyant la présence de deux parlementaires de chaque assemblée en son sein. En outre, nous avons précisé le pouvoir de saisine des assemblées et le délai de réponse de la commission. Sous réserve de ces modifications, le présent projet de loi nous semble constituer un cadre pertinent pour cette politique de développement solidaire, dont la pandémie actuelle nous rappelle, s'il en était besoin, l'absolue nécessité. Les apports issus des nombreux amendements déposés permettront sans nul doute d'aller plus loin et d'améliorer encore le texte. Très bien

d'abord, l'aide au développement « classique », qui vise à lutter contre la pauvreté en fournissant des services essentiels ; ensuite, la défense des droits humains et la bonne gouvernance ; enfin, la préservation des « biens publics mondiaux », comme le climat.

par le Président de la République ou le Premier ministre. La commission a donc prévu la fixation d'un nombre limité d'objectifs figurant au sein du contrat d'objectifs et de moyens (COM), présenté au Parlement avant sa signature. Ce COM rénové

Nous avons enfin adopté en commission de nombreuses améliorations issues de tous les bords politiques. Je citerai le dispositif relatif à la restitution des biens mal acquis, auquel notre collègue Jean-Pierre Sueur, que je salue, a donné la première impulsion,

à savoir les articles 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11 et 13. Annoncé depuis 2018, ce projet de loi constitue un rendez-vous législatif très attendu, bien que repoussé à de nombreuses reprises. Michel Canévet et moi-même, en tant que corapporteurs spéciaux de ce budget pour la commission des finances, l'avions même désigné comme « l'Arlésienne » lors de l'examen du projet d'abord, je tiens à rappeler le constat unanime selon lequel l'intérêt budgétaire de ce texte est très limité. En effet, la trajectoire financière proposée par l'article 1 se contente essentiellement d'entériner les moyens déjà validés par le Parlement. Ainsi, l'évolution pluriannuelle des crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement » prévue par le texte transmis au Sénat commence en 2020 et s'achève en 2022. Cette disposition s'apparente à une transmission avec quelques mois d'avance du projet de loi de finances pour 2022. Aucun des arguments avancés ne justifie cette lacune du texte, d'autant que nous avons adopté récemment la loi de programmation pour la recherche, qui prévoit une trajectoire jusqu'en 2030, ou encore un programme de stabilité jusqu'en 2027. Afin que nous examinions une réelle « loi de programmation », nos deux commissions ont proposé de prolonger la trajectoire des crédits de la mission jusqu'en 2025, en prévoyant une clause de revoyure à mi-parcours. La commission des finances a souhaité proposer une trajectoire visant un double objectif : d'une part, consolider la progression de notre aide publique au développement (APD) pour éviter un nouveau décrochage avec les autres pays développés d'autre part, prévoir une trajectoire crédible et soutenable, compte tenu des contraintes pesant sur nos finances publiques actuellement. Mes chers collègues, je sais que plusieurs autres amendements, tendant à prévoir des hausses plus importantes, ont été déposés. De mon côté, je reste très attaché à l'objectif d'une préservation des moyens de l'APD, mais aussi à la sincérité de la programmation de nos finances publiques. Je vous proposerai, au nom de la commission des finances, un amendement en ce sens, visant à prévoir une hausse annuelle des crédits de 500 millions d'euros après 2022. Initialement, la commission des affaires étrangères a adopté une position différente lors de l'examen du texte. Toutefois, je crois sincèrement qu'un compromis est possible sur ce sujet, et je remercie les rapporteurs des affaires étrangères, nos collègues Hugues Saury et Rachid et Rachid Temal, pour le dialogue constructif que nous avons eu, afin de bâtir une position commune. Par ailleurs, le texte adopté par la commission des affaires étrangères intègre déjà plusieurs amendements sur l'initiative de la commission des finances. visant à améliorer la rédaction du texte, la commission des affaires étrangères a adopté un amendement visant à préciser les modalités de restitution des biens mal acquis. Je remercie à ce titre notre collègue Jean-Pierre Sueur pour les travaux menés sur ce sujet. La commission a également adopté un amendement prévoyant d'avancer la date de remise du rapport annuel, afin que nous puissions disposer de ces informations lors de l'examen de la loi de règlement. Les rapporteurs de la commission des affaires étrangères et moi-même avons également proposé des amendements identiques visant à mettre les dispositions du texte relatives à la nomination des parlementaires au sein des conseils d'administration de l'AFD, d'Expertise France et du Conseil du Conseil national du développement et de la solidarité internationale (CNDSI) en cohérence avec la loi de 2018 sur le sujet. La commission des affaires étrangères a également adopté l'amendement de la commission des finances visant à étoffer l'information du Parlement sur le besoin pluriannuel en fonds propres de l'AFD. En effet, nous devrions être prochainement amenés à nous prononcer sur la question, compte tenu du fait que la recapitalisation prévue par la dernière loi de finances pourrait se révéler insuffisante pour couvrir les besoins en fonds propres de l'Agence dans les prochaines années. Enfin, la commission des affaires étrangères a adopté sur notre initiative un amendement tendant à recentrer les missions de la commission d'évaluation indépendante sur les aides et projets concrets de l'aide publique au développement. Il s'agit de bien séparer

la commission des finances a décidé de vous soumettre deux autres amendements complémentaires. Ils portent respectivement sur la trajectoire des moyens humains de l'État dédiés à la politique de développement et sur la possibilité de débattre en séance publique du rapport annuel prévu à l'article 2. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, 25 ans après la Conférence mondiale de l'ONU sur les femmes à Pékin : où en sont les droits des femmes ? » : telle est la question que se posait la délégation aux droits des femmes, il y a un peu plus d'un an, le 5 mars 2020, à l'occasion d'un colloque organisé pour le vingt-cinquième anniversaire de la Conférence mondiale de Pékin. Si le constat que nous dressions à l'époque était déjà pessimiste sur la réalité de l'avancée des droits des femmes dans certains pays, nous étions encore loin du compte. En effet, la pandémie de covid-19 a exacerbé, à travers le monde, les inégalités et les violences de genre déjà à l'oeuvre avant le début de cette crise sanitaire, économique et sociale. Ainsi, ONU Femmes estime qu'elle pourrait avoir effacé, en une année seulement, les vingt-cinq ans de progrès réalisés en matière d'égalité entre les femmes et les hommes depuis la Conférence mondiale de Pékin. Quelques chiffres me semblent assez marquants pour illustrer le chemin qu'il reste à parcourir : les femmes gagnent encore 20 % de moins que les hommes et elles représentent 70 % des 1,2 milliard de personnes vivant avec moins de un dollar par jour deux tiers des adultes analphabètes sont des femmes et, encore aujourd'hui, plus de 130 millions de filles âgées de 6 à 17 ans ne vont pas à l'école des millions de filles et de femmes sont victimes de violences, de mariages forcés, de mutilations génitales et chaque trimestre de confinement, à l'échelle internationale, engendrerait 15 millions de cas supplémentaires de femmes et de filles exposées aux violences basées sur le genre. Notre délégation travaille depuis de nombreuses années sur les droits des femmes et des filles dans le monde. Tous nos travaux nous ont confortés dans cette conviction l'égalité des sexes et l'autonomisation économique et sociale des femmes constituent le socle essentiel d'un développement durable dans tous les pays en voie de développement. C'est pourquoi il nous paraît essentiel, aujourd'hui, d'orienter au mieux le financement de l'aide publique au développement vers des projets favorables au renforcement des droits des femmes et à l'égalité de genre. En la matière, la France soutient de longue date les engagements internationaux conclus, dans le cadre de l'ONU notamment, en faveur des droits des femmes, engagements qu'elle défend à l'échelle internationale dans ses relations bilatérales comme dans les enceintes multilatérales. À cet égard, je citerai l'Agenda 2030 pour le développement durable, adopté par les 193 membres de l'ONU en 2015, qui fixe 17 objectifs de développement durable (ODD), parmi lesquels l'ODD 5 qui vise à « parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ». La France souscrit également aux critères de marquage « genre » des projets de développement, définis par le Comité d'aide au développement de l'OCDE. D'importantes avancées sont intervenues récemment pour mieux orienter les financements de la politique de développement vers des projets favorables à l'égalité entre les femmes Pour autant, nous devons rester vigilants sur la mise en oeuvre de cette politique comme sur les moyens, humains et financiers, qui lui sont alloués. C'est dans ce contexte qu'intervient l'examen par notre assemblée du projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Du point de vue de l'intégration du genre comme priorité de la solidarité internationale, on peut se féliciter du travail accompli par nos collègues députés lors de l'examen du texte. Ils ont en effet inséré dans le projet de loi un nouvel article 1 A, qui inscrit directement dans la loi les grands objectifs de la politique de développement. Cet article précise notamment que, dans le cadre de la diplomatie féministe de la France, la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales a pour objectif transversal la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes.

la délégation aux droits des femmes a formulé neuf recommandations permettant de mieux intégrer l'égalité de genre au sein de notre politique d'aide publique au développement, de sa conception à sa mise en oeuvre sur le terrain. Nous estimons que, si ces recommandations sont appliquées, elles permettront à la France de se donner les moyens de ses ambitions en matière de diplomatie féministe. Nous avons déposé des amendements en ce sens. collègue. En cette période de crise mondiale sans précédent, nous nous devons de protéger encore davantage toutes les femmes et les filles victimes d'inégalités et de violences à travers le monde.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis pour examiner un projet de loi très attendu, qui prend une résonance toute particulière avec la crise liée à la pandémie de covid. Cette crise frappe plus durement les pays pauvres et fragiles.

Les progrès accomplis ces dernières décennies en matière de lutte contre la pauvreté, de santé et d'éducation sont dangereusement remis en cause. Face à ce constat alarmant,

Un surcroît d'ambition et de mobilisation est d'autant plus nécessaire qu'un retard dans la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 avait été constaté. Avec le texte ambitieux dont nous sommes saisis,

Notre pays est par ailleurs pleinement mobilisé pour aider l'Afrique à sortir de la pauvreté, ce qui est l'une de nos priorités, en concentrant les moyens de l'APD sur 19 pays prioritaires, dont 18 pays d'Afrique subsaharienne et en particulier 5 du Sahel. Sahel. Aussi le Président de la République pourra-t-il faire des annonces lors du Sommet sur le financement des économies d'Afrique subsaharienne prévu le 18 mai prochain. L'adoption unanime du projet de loi à l'Assemblée nationale témoigne du caractère consensuel de la réforme proposée par le Gouvernement. Je me félicite de l'état d'esprit constructif dans lequel notre commission a mené ses travaux, a mené ses travaux, de façon convaincante et à vive allure. Je suis convaincu qu'un même état d'esprit nous animera d'ici à la fin de la discussion du texte en séance publique. Je remercie le président Cambon, les rapporteurs et tous les collègues qui ont bien voulu travailler avec nous. Pour ce qui concerne la programmation financière, il reste quelques divergences.

tous les moyens dont elle dispose pour atteindre l'objectif de 0,7 % du RNB consacré à l'APD en 2025. J'espère qu'une rédaction de compromis pourra être trouvée. Par ailleurs, tout en me réjouissant de la volonté de nos rapporteurs de consacrer à l'APD 60 % du produit de la TTF, je m'interroge sur l'opportunité d'abonder un instrument extrabudgétaire, le qui échappe au contrôle du Parlement et a longtemps servi à compenser la baisse des crédits de la mission « Aide publique au développement ». S'agissant de la commission indépendante d'évaluation, le groupe RDPI a déposé plusieurs amendements visant à assurer

doivent-ils siéger au sein de la commission, sachant que l'Assemblée nationale et le Sénat disposent de leur propre capacité d'évaluation et qu'ils seront destinataires des rapports ? les personnalités qualifiées doivent-elles être désignées par le Gouvernement, qui assure le pilotage de la politique d'APD ? Troisièmement, quel rôle la Cour des comptes et son premier président doivent-ils jouer ? Nous devrons en outre veiller à ce que la commission puisse se pencher sur la question du détournement de l'APD. Ce phénomène est difficile à évaluer. La Banque mondiale s'y est récemment essayée. En ce qui concerne les 22 pays les plus dépendants de son aide, elle estime à au moins 5 % la part des flux détournés vers des paradis fiscaux. Cela m'amène à évoquer la question des biens dits « mal acquis ». Le procès en appel de l'oncle de Bachar el-Assad pour blanchiment de détournement de fonds publics montre, s'il en était encore besoin, combien il est nécessaire de créer un dispositif permettant la restitution, au plus près des populations concernés. Pas moins de 500 millions d'euros de biens et de valeurs auraient été saisis en France ces dernières années. Le dispositif prévu à l'article 1 s'inspire très largement de loi de notre collègue Jean-Pierre Sueur, que je tiens à saluer et que nous avons suivi au travers de la rédaction de nos amendements. Une autre avancée majeure est l'intégration, réclamée

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est peu de dire que nous attendions, sous le sceau de l'urgence, ce projet de loi de programmation pour l'aide Face à l'ampleur des inégalités sociales et économiques mondiales, face aux déstabilisations qu'elles entraînent dans nombre d'États et de régions du monde, face à la pandémie aujourd'hui, au danger climatique, aux crises de plus en plus nombreuses, le développement solidaire de l'humanité n'est plus une option c'est devenu la condition première de la sécurité humaine collective. Le droit à un développement humain digne est le premier des biens communs à promouvoir. Nous en sommes loin ! La France doit changer d'échelle en matière d'APD et redéfinir le contenu de son aide. Les objectifs justement rappelés, un ajout de l'Assemblée nationale, en tête du projet de loi- éradication de la pauvreté, lutte contre les inégalités, promotion des droits humains, de l'éducation et de la santé, des droits des femmes, protection des biens publics mondiaux -, doivent guider toute notre action et non une logique d'influence au service d'une puissance réservée à un petit club de nations les plus riches et de quelques grands groupes privés. grands groupes privés. C'est au service du développement de tous les peuples que le rayonnement de la France peut prendre du sens, et non au service d'une logique de concurrence et de puissance de plus en plus contestée et contestable. Le débat sur la levée des brevets des vaccins illustre parfaitement ces deux logiques. Considérer d'abord l'APD à l'aune, comme vous l'avez déclaré, monsieur le ministre, des « bénéfices à en attendre pour notre pays », ce serait continuer à rater la cible d'une politique solidaire internationale à la hauteur. À son arrivée au Sénat, ce texte n'avait de programmation que le nom. La commission a faiblement corrigé cela avec la programmation des crédits budgétaires jusqu'en 2025. Nous proposons une autre ambition : premièrement, en inscrivant enfin et clairement dans la loi l'objectif contraignant des 0,7 %, auquel la France se dérobe depuis des années deuxièmement, en fixant les objectifs chiffrés qui vont avec car, nous le savons, les taux ne suffisent pas ; troisièmement, en pérennisant cette ambition jusqu'en 2030. Membre du Conseil de sécurité de l'ONU, la France ne peut pas décemment continuer à tourner le dos à ces objectifs fixés par l'Assemblée générale des Nations unies en 1971

La pandémie et ses terribles conséquences appellent un engagement massif contre les inégalités mondiales, pour le développement et la sécurité de tous. C'est le moment de garantir dans la durée une véritable ambition. Sans cela, le tournant dont vous parlez ne sera que belles paroles. Pour financer cette ambition, il faut non seulement garantir nos choix budgétaires, mais nous vous proposerons également d'augmenter l'assiette, le rendement et l'affectation de la taxe sur les transactions financières. Car la financiarisation délirante du monde capitaliste, à l'origine du krach mondial de 2008, est une indécence chaque jour lancée à la face des plus pauvres de la planète. Garantir une nouvelle ambition, c'est aussi réorienter notre aide en profondeur avancés (PMA), aux services sociaux de base, à l'émancipation des femmes, aux dons et non aux prêts. Ces objectifs doivent être gravés dans le marbre avec des cibles chiffrées. Enfin, et j'ai envie de dire qu'il s'agit en fait de l'essentiel, il convient de changer en profondeur la philosophie de notre aide, pour la tourner résolument vers la construction des bases solides d'un développement propre des pays destinataires et la dégager de toutes les logiques de pillage qui persistent encore largement. Nos amendements iront dans ce sens, privé (ISP) et les contrats de désendettement, lesquels doivent être mis en cause et sortis des comptes de l'APD, car ils maintiennent les pays concernés dans la dépendance financière au lieu de les en dégager. Nous devons également consacrer des fonds importants à la construction de recettes fiscales pérennes et solides pour les pays bénéficiaires, comme le FMI commence même à le prôner. Enfin, la cohérence de toutes nos politiques doit être recherchée. Car à quoi sert d'aider d'une main si nous prenons de l'autre autant, et trop souvent plus ? Accords commerciaux et libre-échange, lutte contre le changement climatique, conventions fiscales, relations monétaires, conditions d'engagements léonines des grands groupes français tout doit être réexaminé si nous voulons que la cohérence en faveur du développement entre dans la réalité. Nous proposons à cette fin qu'un rapporteur spécial suive dans chaque assemblée du Parlement la mise en oeuvre de cette cohérence transversale. Pour toutes ces raisons, nous soutenons, avec des suggestions d'amélioration, l'instauration d'un rapport et d'un débat annuel ainsi que la création d'une commission indépendante d'évaluation.

monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui le projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Ce texte, très attendu, est notamment la concrétisation de l'engagement du Président de la République, pris au début de son mandat et rappelé lors de son discours à l'université de Ouagadougou,

Elle a exacerbé des inégalités déjà existantes et en a créé de nouvelles. Au-delà de la crise sanitaire mondiale que nous traversons, le déploiement de l'APD française s'inscrit dans un contexte géopolitique marqué par l'urgence climatique, mais aussi par la persistance des crises, l'aggravation des inégalités mondiales, la résurgence de logiques de puissances nationales affaiblissant le multilatéralisme, les guerres persistantes et les difficultés certaines à faire respecter les droits humains fondamentaux. Les ambitions, les outils et les moyens de la politique de développement solidaire ayant eux aussi évolué, il était nécessaire que nous puissions débattre sur ces sujets.

Je pense également à l'amélioration de la redevabilité de la politique de développement solidaire, un rapport annuel du Gouvernement au Parlement, qui comportera toutes les informations nécessaires à la compréhension globale des actions menées au cours de l'année qui précède et où sera notamment mentionnée la liste des pays dans lesquels intervient l'AFD. Cette mention nous permettra, lors du débat qui suivra la remise de ce rapport, d'échanger sur les financements accordés à certains pays émergents. La création d'une commission indépendante d'évaluation de la politique de développement solidaire et la transformation d'Expertise France en société par actions simplifiée au sein du groupe AFD sont également des avancées auxquelles nous souscrivons. Cependant, si ces avancées doivent être saluées, certaines dispositions nous semblent trop timides. La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a contribué à clarifier le texte, plusieurs modifications, et, à cette occasion, je souhaite remercier les corapporteurs de la qualité de leurs travaux. La priorisation des objectifs était nécessaire pour une meilleure lisibilité des politiques de développement, et je salue l'inscription de la protection de la planète comme l'un d'entre eux. En effet, la crise sanitaire due au covid ne doit pas placer la situation d'urgence climatique au second plan. La commission a également proposé une véritable programmation jusqu'en 2025, rendu la taxe sur les transactions financières à sa vocation première, amélioré l'information du Parlement et renforcé la tutelle de l'État sur l'AFD. Enfin, elle a oeuvré pour que la part de dons de l'APD soit renforcée en fixant un objectif de 65 % de dons, contre 59 % actuellement. Il nous semble que le texte proposé par notre commission est équilibré, mais nous insisterons sur quelques points. Nous soutiendrons plusieurs amendements afin de défendre l'usage du français dans les instances internationales, la promotion de son apprentissage et l'aiguillage de financements de l'AFD vers les établissements enseignant notre langue. Nous souhaitons également que le français soit la langue de travail de l'AFD. Il nous a semblé que les territoires d'outre-mer n'étaient pas reconnus à leur juste valeur ; aussi, nous vous proposerons un amendement visant à clarifier leur rôle dans le cadre de la politique de développement solidaire, afin d'en faire des territoires relais, essentiels dans leur environnement régional. Nous proposerons également un dispositif alternatif à celui de l'article 9, en soutenant l'amendement de notre collègue Michel Canévet. Le Parlement contrôle et évalue, en vertu de son rôle constitutionnel, les politiques d'aides publiques. vise donc à regrouper et à centraliser les activités de contrôle de la politique française de développement, tout en les élargissant au sein de cette nouvelle commission indépendante. Les différents groupes parlementaires d'amitié seraient en particulier associés aux travaux de la commission, en apportant leur éclairage et leur évaluation sur leur zone de compétence. Un autre amendement tend à approfondir cette participation des groupes d'amitié à la politique de développement, en les associant aux travaux des conseils locaux de développement, autre nouveauté de ce texte. Enfin, nous soutiendrons, par un amendement de notre collègue Olivier Cadic, nos entrepreneurs français à l'étranger, qui contribuent directement à la création de richesse dans les pays dans lesquels ils s'implantent. au droit local, ces entrepreneurs français à l'étranger ne bénéficient d'aucune aide française dans le cadre de la pandémie ou lors de catastrophes naturelles, par exemple. Ouvrir le dispositif de garantie et d'aides à l'ensemble des entrepreneurs français à l'étranger dans le besoin permettrait d'épauler un partenaire majeur de l'aide publique au développement lorsqu'ils sont en difficulté. À l'heure actuelle, l'actualité mondiale nous montre plus que jamais à quel point l'aide publique au développement est cruciale. Plusieurs pays, plusieurs régions du monde, sont en proie à des déséquilibres qui laissent craindre, dans un futur proche, l'émergence de situations contraires à nos intérêts. L'APD, levier puissant de notre diplomatie et de notre rayonnement, doit répondre aux défis communs par la pérennisation de la solidarité internationale. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en ces temps de crise, la tentation est grande pour les pays de faire l'impasse sur l'aide au développement. Alors que la France fait face à de nombreuses difficultés et que les conséquences économiques de la crise que nous traversons sont loin d'être derrière nous, certains pourraient s'interroger sur l'opportunité de consacrer une part de notre budget au développement d'autres pays. Nous sommes cependant convaincus que céder à la tentation du repli sur soi serait une erreur. L'interdépendance des économies est une réalité. Aider au développement des autres, c'est contribuer au sien. Par ailleurs, le développement est un moyen efficace de prévenir l'apparition, dans des zones défavorisées, de conflits dont les conséquences s'étendent bien souvent jusqu'en France. Nous nous félicitons donc de ce que le Gouvernement soumette à l'examen du Parlement un projet de loi de programmation de l'aide française au développement. Ce texte fixe les objectifs de dépense en la matière. En 2022, la barre des 0,55 % du RNB devrait être franchie. En 2025, c'est le seuil de 0,7 %, préconisé par les Nations unies, qui devrait être atteint. Nous nous félicitons en outre de ce que les fonds consacrés au soutien de l'action extérieure des collectivités atteindront en 2022 le double du montant de 2017. L'augmentation des moyens destinés à l'aide au développement devrait permettre à la France de conserver son rang, dans un domaine où d'autres puissances sont de plus en plus présentes. Cette loi ne prévoit pas seulement de fixer les niveaux de dépenses. Elle tend également à mieux définir le cadre de la politique française d'aide au développement. Un tel encadrement est nécessaire pour que les montants engagés puissent produire tous leurs effets. La commission des affaires étrangères a tenu à préciser encore la programmation de l'aide. Elle s'est notamment penchée sur le pilotage de l'aide française. Plusieurs points restaient à améliorer pour que notre politique atteigne pleinement les objectifs qu'elle se fixe. Par le passé, la France a en effet pu consacrer des fonds à des pays qui paraissaient assez peu prioritaires. La forme que revêtait cette aide n'a pas non plus toujours permis aux pays destinataires de voir leur situation s'améliorer réellement. Dans cette perspective, nous soutenons un meilleur encadrement de l'AFD, ainsi que la détermination d'objectifs clairs dans la loi de programmation. Le texte réserve une place particulière à la forme que doit revêtir notre aide : davantage d'aide bilatérale et plus de dons que de prêts. Une part substantielle devra en outre être consacrée à des pays prioritaires dûment Les États concernés font partie des pays les moins avancés. Plusieurs d'entre eux font actuellement face à une situation sécuritaire très préoccupante, notamment les pays du G5 Sahel, ce qui rend notre aide encore plus nécessaire. L'inscription de ces évolutions dans la loi et le renforcement de la composante bilatérale amélioreront l'efficacité de l'aide française à destination des pays qui en ont le plus besoin. Le texte a également repris l'objectif de mieux associer la société civile à ce processus. Cette dernière constitue en effet un acteur important et innovant du développement des pays destinataires. Mieux l'impliquer dans notre politique permet aussi de diversifier les vecteurs de notre aide et de nous assurer qu'elle bénéficie effectivement à la population. La France fait partie des plus grands contributeurs mondiaux de l'aide au développement. Nous devons nous assurer que notre aide parvient là où elle est la plus nécessaire, mais aussi qu'elle produit les effets escomptés. À cet égard, nous saluons la création de la commission indépendante d'évaluation de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

et un ans que la France tente péniblement de tenir cette promesse, l'extraordinaire explosion de la richesse mondiale a permis de faire reculer l'extrême pauvreté. Toutefois, elle n'a nullement réduit les inégalités entre les êtres humains ou entre les pays riches et les pays pauvres. Aujourd'hui encore, quelque vingt pays concentrent 90 % du PIB mondial. Aujourd'hui encore, 690 millions de personnes, soit près de 10 % de l'humanité, souffrent de la faim. Et ce chiffre augmente, pour la quatrième année consécutive, sur fond de guerres, de catastrophes climatiques, de pandémie et d'accroissement des inégalités. L'ONU estime que, faute d'action suffisante, le nombre de personnes souffrant de la faim pourrait quasiment doubler d'ici à 2080. Plus que jamais, l'effort de solidarité internationale doit être décuplé. Naturellement, l'APD n'est que le pansement sur la jambe de bois du système capitaliste. Elle ne permet pas de lutter contre les effets délétères du changement climatique et de la prédation des pays riches sur les ressources des pays en développement. Elle ne permet pas non plus de lever les brevets des vaccins et d'assurer l'immunité rapide des populations des pays pauvres face au covid-19. Elle ne permet pas, enfin, d'assurer une meilleure répartition des richesses mondiales ou de prévenir les velléités belliqueuses des Nations. Toutefois, faute de grand soir, faute de révolution écologiste, il est indispensable d'agir sans attendre pour venir en aide à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Le présent projet de loi a vocation à servir cette ambition. Il est désormais porteur d'une trajectoire budgétaire renforcée, ainsi que de l'esquisse d'un chemin pour parvenir enfin, en 2025, à une part de 0,7 % du RNB consacrée à l'APD ; il prévoit il prévoit aussi une timide augmentation des dons, de l'aide bilatérale et du partenariat avec les organisations de la société civile. Notre responsabilité est de consolider ces acquis en s'assurant d'une priorité absolue consacrée aux PMA ; d'un d'un renforcement net de la part des dons, plutôt que des prêts, dans le volume de l'APD française ; de l'accroissement des moyens transitant par les organisations de la société civile ; de l'augmentation, au moins au niveau de la moyenne de l'OCDE, des programmes ayant pour objectif l'égalité entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons du renforcement des financements mobilisés pour la protection de la biodiversité ; enfin, de la transparence sur les données de l'APD française. Nous vous proposerons à cet effet des amendements visant à renforcer l'ambition de cet article 1. L'Assemblée nationale a fait le choix judicieux d'inscrire dans le corps de la loi les principaux objectifs de la politique de développement française. De l'éradication de la pauvreté à la préservation des biens publics mondiaux, de la défense des droits humains à la promotion de l'accord de Paris, de la diplomatie féministe au renforcement de la démocratie : nous nous retrouvons dans cette feuille de route exigeante. Il nous semble néanmoins nécessaire de la compléter, pour accroître l'attention portée à certains publics fragiles, mais également de renforcer l'indispensable cohérence entre la politique française de développement et les autres politiques publiques. En effet, trop souvent, nous défaisons d'une main ce que nous construisons de l'autre. Prenez le projet Feronia : de 2012 à 2020, Proparco, filiale de l'AFD, a financé un funeste projet de production d'huile de palme sur une superficie équivalant à celle de la Belgique, entraînant des accaparements fonciers, écocides, des violations des droits humains et même des meurtres ... Feronia n'est pas une exception ; les projets agricoles néfastes pour l'environnement et les économies locales sont, hélas, encore fréquents dans les financements français. La restructuration de l'AFD, le renforcement de la tutelle de l'État et la mise en place d'une commission d'évaluation indépendante qui sont prévus par le texte permettront, je l'espère, de lutter contre ces graves violations de nos engagements. Nous aurons le regret, toutefois, que l'intégration d'Expertise France à l'AFD se rapproche d'une simple juxtaposition et ne garantisse pas à nos experts de la coopération technique internationale le statut des personnels de l'AFD, fragilisant du même coup la cohésion du groupe AFD et la qualité de notre aide. Monsieur le ministre, un tiens valant toujours mieux que deux tu l'auras, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires se prononcera, non sans exigence, non sans espoir, en faveur de ce projet de loi.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les efforts de la communauté internationale, déployés depuis des décennies dans un cadre de coopération sans cesse renforcé, ont permis de faire reculer l'extrême pauvreté. Cependant, près de la moitié des habitants de la planète sont toujours en situation de grande fragilité, une réalité que la pandémie de covid pourrait aggraver. Or nous savons bien que la misère est source de conflictualité dans de nombreuses régions du monde. Il est ainsi peu surprenant de voir le terrorisme islamiste s'enkyster au Sahel, où se concentre la majorité des PMA, les pays les moins avancés. Si l'aide au développement a par essence une vocation humanitaire, je soulignerai qu'elle est aussi un gage de stabilité politique pour les pays aidés et, par ricochet, pour la sécurité de tous. Pour le dire autrement, je citerai François Mitterrand. Quelle référence ! Mais

La France doit donc continuer plus que jamais à tenir son rôle de grand contributeur de l'aide mondiale. En 2017, le Président de la République a fixé un cap : porter l'aide publique de la France à 0,55 % de son revenu national brut. Nous nous en réjouissons.

et le RDSE se réjouit des grandes orientations proposées. Je ne reviendrai pas en détail sur la question de la trajectoire financière, que les deux commissions ont consolidée en sécurisant les montants des crédits jusqu'en 2025, ce qui était en effet nécessaire. Je salue toutefois une autre initiative de notre collègue rapporteur pour avis et président du RDSE, Jean-Claude Requier, celle qui vise à compléter le document de politique transversale avec une évaluation pluriannuelle des besoins en fonds propres de l'AFD, une dimension qui manquait en effet à cette programmation. Mes chers collègues, en marge des moyens budgétaires, que devons-nous attendre de notre politique de développement solidaire ? À l'évidence, de la cohérence et de l'efficacité. La cohérence, c'est faire converger tous les outils dans la même direction, ce à quoi répond l'article 3, en intégrant les ODD comme cadre de référence de notre politique, en écho à nos engagements aux Nations unies. La cohérence, c'est aussi prendre en compte les stratégies de développement des pays aidés et les besoins de la population, comme le rappelle le nouveau cadre de partenariat global, le CPG. Enfin, au travers de l'article 2, il est exigé que nos politiques publiques soient cohérentes avec celle de l'aide au développement. Dans cet esprit, en commission, nous avons souhaité inscrire dans la loi le principe de coordination entre les acteurs militaires et les acteurs de l'aide au développement au Sahel. C'est en effet important. S'agissant de l'efficacité de l'aide au développement, celle-ci repose à mon sens sur plusieurs piliers. J'en citerai quelques-uns. Mon groupe approuve la philosophie globale des articles consolidant le pilotage de l'APD, que ce soit le rapprochement d'Expertise France avec l'AFD, le renforcement le renforcement de la tutelle de l'État sur l'opérateur, ou encore l'affirmation de l'autorité du chef de mission diplomatique sur les agences de l'opérateur à l'étranger. L'État reprend la main On peut le concevoir au regard des sommes de plus en plus importantes engagées par l'AFD. L'efficacité, c'est aussi choisir les bonnes priorités géographiques, c'est-à-dire mettre les moyens au bon endroit. L'Afrique est une nouvelle fois désignée comme prioritaire, une exigence formulée depuis longtemps, mais qui ne se traduit pas suffisamment dans les faits. Pourtant, le continent africain est celui de tous les défis : un défi démographique, avec 2 milliards d'habitants attendus à l'horizon de 2050, un défi climatique, à l'évidence, un défi sanitaire, hier avec le virus Ebola, aujourd'hui avec l'accès aux vaccins contre le covid, et, enfin, un défi sécuritaire, que j'ai déjà évoqué. La concentration de notre effort sur l'Afrique est dans ces conditions fondamentale. Mes chers collègues, si j'avais davantage de temps, j'insisterais également sur les impératifs d'évaluation, de transparence, de redevabilité et de perception de la part des populations. Il est positif que ces objectifs soient consolidés, parce que notre politique de développement doit être exemplaire dans toutes ses dimensions,

monsieur le ministre, mes chers collègues, enfin ! Enfin, nous abordons, avec beaucoup de retard, l'examen de ce qui devait être l'une des grandes priorités du quinquennat. Ce retard a forcément des conséquences sur une programmation 2020-2025 qui commence en 2021 et se termine en 2022.

progresser. C'est possible sur le ciblage géographique. La qualité de l'APD dans la lutte contre l'extrême pauvreté va de pair avec un ciblage efficace vers les pays et les populations qui en ont le plus besoin. l'aide française souffre d'une forte dispersion. Les 19 pays dits « prioritaires » ne reçoivent que 13 % de l'aide. La loi fixe des priorités qui ne se traduisent pas dans les faits. C'est la même chose pour les pays du G5 Sahel. Tous, nous connaissons les racines du mal : c'est la misère qui pousse les populations dans les bras des terroristes, c'est la colère des peuples qui s'élève contre la mal-gouvernance et la corruption et qui, en juin 2020, a provoqué la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta au Mali. Cette colère se porte malheureusement aujourd'hui aussi contre la présence des forces françaises dans la région. Nos soldats nous le disent, l'autre volet de la lutte contre le terrorisme, c'est une politique de développement volontariste au Sahel. Je voudrais souligner ici l'une des grandes avancées portées par les socialistes, soutenue par les corapporteurs et, j'y insiste, par l'ensemble des membres de la commission : consacrer un article dédié aux organisations de la société civile, reconnaissance formelle de leur rôle dans la politique d'aide au développement. Cette dimension partenariale, dans l'élaboration comme dans la mise en oeuvre de cette politique, me paraît indispensable dans un texte de loi. Si le Gouvernement ne nous suivait pas sur ce point, ce serait un très mauvais signe en direction de celles et de ceux qui sont engagés au quotidien sur le terrain. Tout aussi remarquable est l'avancée sur les biens mal acquis. Grâce à l'action de Jean-Pierre Sueur, sénateur socialiste et questeur de cette institution, et, je dois le dire, grâce au soutien de l'ensemble de cette assemblée, un travail a pu être engagé, qui a abouti à un accord avec le Gouvernement. Les fonds provenant de la confiscation des biens mobiliers et immobiliers que s'approprient les brigands de tous bords seront directement reversés aux populations spoliées. Un mécanisme a été trouvé. Félicitons-nous de cette avancée et continuons de lutter contre la corruption internationale et les paradis fiscaux. Posons le principe d'un devoir de vigilance à l'égard de nos entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. L'enregistrement des naissances doit aussi figurer au premier rang de nos objectifs. 237 millions d'enfants n'ont pas d'acte de naissance : ils n'existent pas. On ne peut donc pas les protéger contre la prostitution, l'esclavage, le travail forcé, l'enrôlement comme enfants-soldats ... Ils deviendront des adultes invisibles. La France doit contribuer au fonds qui est en train de se mettre en place en faveur de l'enregistrement des naissances, sous l'égide des Nations unies. Nous vous le demandons instamment, monsieur le ministre. L'urgence d'une vaccination mondiale est réelle. Si une vaccination massive n'intervient pas d'ici à un an, la situation sanitaire dans les pays les plus pauvres deviendra incontrôlable. Le mécanisme de solidarité Covax n'a pas produit les effets escomptés. Il est temps d'aller plus loin et de supprimer tous les obstacles juridiques liés aux droits exclusifs de la propriété intellectuelle, qui limite artificiellement la production massive de vaccins anti-covid. Il aura fallu la déclaration de Joe Biden pour qu'Emmanuel Macron emboîte le pas. Je ne doute pas que l'ensemble du Gouvernement s'alignera désormais derrière la nouvelle position du Président de la République, et que, à rebours de vos déclarations passées ici même, monsieur le ministre, vous soutiendrez nos amendements en faveur de la levée des brevets contre la covid-19. évoquant le pilotage politique. Il est impossible de savoir qui fait réellement quoi, comme je l'avais déjà souligné. Or les Français n'y verront toujours pas clair sur la politique d'aide au développement de la France : loin de clarifier la gouvernance, cette loi se contente de dessiner les contours flous d'un pouvoir plus que jamais présidentiel. De nouveau, la verticalité s'exprime, par la création du conseil du développement auprès du Président de la République. Nous n'en voyons pas l'intérêt. En revanche, il y a un grand absent : c'est le ministre de la coopération.

Plus que jamais, la politique de développement doit être un phare pour la France. Dans un monde bouleversé, fracturé, en proie à de multiples crises et maintenant malade, c'est notre devoir, à nous tous ici, de contribuer à faire reculer la misère. Un devoir moral, éthique,

Enfin, nous y voilà, monsieur le ministre ! Du temps nous a été donné pour examiner ce projet de loi relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales,

Depuis plusieurs années, nous observons avec une certaine inquiétude un monde plus chaotique, une montée des égoïsmes nationaux, une expansion du terrorisme, un changement climatique menaçant. Dans ce contexte, la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales a un rôle essentiel à jouer. Il ne s'agit pas là d'une posture empreinte d'un quelconque angélisme, car cette politique constitue un moyen d'influence et d'affirmation incontournable de la France sur la scène internationale. Lorsqu'elle est à la hauteur des enjeux, cette politique peut contribuer à renforcer la crédibilité de notre action diplomatique. Dans des circonstances où notre pays est fortement engagé sur le plan militaire, en particulier pour lutter contre le terrorisme, l'aide au développement doit aussi combattre l'extrême pauvreté, véritable terreau

À défaut, nous pourrions décupler les effectifs de Barkhane sans obtenir aucun succès durable. Ainsi, en 2019, nous avons dépensé environ trois fois plus pour notre action militaire qu'en APD bilatérale pour l'ensemble des 5 pays du Sahel. C'est bien en luttant contre la pauvreté et en construisant des sociétés solides, où les citoyens, en particulier les jeunes, retrouvent des perspectives d'éducation, de santé et de travail, que nous sortirons de cette crise et que nous en éviterons d'autres. Permettez-moi, à présent, de rappeler les grandes priorités qui nous ont guidés dans l'examen du texte en commission. Premièrement, l'aide publique au développement ne doit jamais perdre de vue nos trois grandes priorités : nourrir, soigner et former. Notre commission a reformulé dans cet esprit, à la fois les grands objectifs de cette politique et les missions de l'Agence française de développement. Viennent ensuite, bien sûr, les grands objectifs de nature transversale : la protection du climat et de la biodiversité, l'égalité femmes-hommes et la bonne gouvernance. Deuxièmement, nous souhaitons rééquilibrer notre aide publique au développement en augmentant la part des dons par rapport aux prêts, celle du bilatéral par rapport au multilatéral, enfin, la part consacrée aux pays les plus pauvres par rapport à celle qui bénéficie aux pays à revenu intermédiaire. C'est une nécessité pour mieux cibler les 19 pays prioritaires de l'aide française. Faisons une comparaison avec le Royaume-Uni, qui, certes, a récemment réduit son effort. En 2018, quelque 11 pays africains ont reçu chacun plus de 100 millions de dollars d'APD des Britanniques et 5 pays chacun plus de 200 millions La même année, seuls 2 pays recevaient plus de 100 millions de dollars de la part de la France, dont 1 seul pays prioritaire, le Sénégal. Les nouveaux critères fixés par notre commission doivent ainsi nous permettre de concentrer davantage notre effort, pour obtenir un réel impact. Troisièmement, au sein de cette loi dite « d'orientation et de programmation », nous avons eu un peu de mal à trouver cette programmation. De report en report, le texte ne programme plus que pour l'année 2022, à quelques mois du projet de loi de finances.

plusieurs lois de programmation récentes vont au-delà de la présente législature, qu'il s'agisse de la recherche ou de la fameuse loi de programmation militaire. Nous espérons ainsi sanctuariser des moyens annuels supplémentaires, qui permettront notamment de soutenir des pays durement touchés par la crise économique consécutive à la crise sanitaire. Quatrièmement, nous avons mis l'accent sur le pilotage et l'évaluation, est un de nos chevaux de bataille depuis bien longtemps. La politique de développement solidaire pèse plus de 12 milliards d'euros, mes chers collègues, et bien davantage si l'on tient compte de l'ensemble des engagements en prêts de l'AFD, sans parler des apports réguliers de fonds propres à l'agence. De tels montants rendent nécessaires un pilotage efficace, davantage de transparence et un meilleur contrôle démocratique. À cet égard, nous saluons vos efforts, monsieur le ministre, pour améliorer le pilotage de cette politique et l'exercice de la tutelle sur l'Agence française de développement. C'est d'autant plus nécessaire que le texte prévoit l'intégration à terme d'Expertise France au sein de l'AFD, conférant ainsi à l'agence une présence encore plus dominante dans le paysage de l'APD française. Nous saluons également la création du conseil local de développement, dirigé par un ambassadeur. En améliorant la cohérence entre politique de développement et politique diplomatique, il pourra nous épargner bien des erreurs d'appréciation, liées à une approche trop centralisée. Récemment encore, le président Larcher et moi-même avons eu un aperçu du chemin qui reste à parcourir dans ce domaine, en constatant un manque total de coordination entre le centre de crise du Quai d'Orsay et notre ambassade en Arménie. Celle-ci a en effet vu arriver des tonnes de pâtes et de couches-culottes qu'elle n'avait jamais demandées. Il faudra donc faire vivre ce nouveau conseil local, pour donner à l'ambassadeur le rôle de chef d'orchestre qui lui revient. Par ailleurs, le contrôle démocratique sera renforcé par la création de la nouvelle commission indépendante d'évaluation, que nous appelions depuis longtemps de nos voeux. Nous avons souhaité préciser sa composition en prévoyant notamment la présence de quatre parlementaires. porteront au sein de cette nouvelle instance une exigence de lisibilité, d'efficacité et de démocratie. Le Gouvernement doit s'appuyer sur le Parlement, et non craindre son regard ; je sais que tel est votre sentiment, monsieur le ministre. Nous aurions toutefois souhaité aller plus loin dans l'amélioration du pilotage. En commission, nous avons renforcé le rôle du ministre chargé du développement. La politique de développement solidaire étant essentielle au rayonnement et à la promotion des intérêts de la France, il serait toutefois préférable, selon nous, qu'elle soit incarnée, à vos côtés, par un ministre ou un secrétaire d'État dédié. Peut-être une prochaine législature le permettra-t-elle. Je souhaite, pour finir, souligner que l'examen du projet de loi en commission, sous l'égide de nos excellents rapporteurs Hugues Saury et Rachid Temal, a eu lieu dans une atmosphère consensuelle. Nous avons adopté de nombreux amendements qui visaient à apporter au texte initial

ce sujet en valant vraiment la peine. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous le savons tous, la France rayonne à travers le monde par son histoire, par son message et par ses valeurs.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, « il y a toujours un avenir pour ceux qui pensent à l'avenir Alors que nous fêtions hier les quarante ans de l'accession au pouvoir de François Mitterrand, cette phrase que je lui emprunte nous rappelle l'impérieuse nécessité de penser le futur afin de nous garantir un avenir. La pandémie nous montre cruellement que, dans ce monde globalisé, personne ne sera en sécurité tant que tout le monde ne le sera pas collectivement. En matière d'aide publique au développement, la maxime de notre action doit être l'intérêt commun. Nous déplorons le manque d'ambition de la trajectoire financière proposée dans ce texte. Refuser de respecter l'engagement pris en 1970 de consacrer à l'aide publique au développement 0,7 % du revenu national brut nous paraît complètement anachronique, voire hors sol. Nous libérons 300 milliards d'euros dans un plan de relance sur un an et nous serions incapables de libérer 524 millions d'euros supplémentaires sur cinq ans

Force est de constater que les robinets sont grands ouverts, mais coulent dans le même évier. En commençant en 2020 et en s'arrêtant en 2022, cette loi de programmation n'a de programmatique que le nom. Quand on pense des politiques d'aide au développement, il est impérieux de les inscrire dans la durée, car ce sont des projets non pas de court terme, mais de long terme, et les pays avec lesquels nous travaillons doivent pouvoir les anticiper. Le FMI estime que les épidémies ont un effet pacificateur à court terme, car elles renforcent la cohésion sociale et la solidarité, qui sont des éléments propres à tout événement catastrophique. En ce sens, la politisation extrême de la pandémie est un élément incontournable des relations internationales depuis un an, bien alimentée par la rivalité sino-américaine qui n'est même plus voilée. Dans ce contexte, chaque pays tient à répondre présent, la Chine par le biais des masques, l'Allemagne par celui des respirateurs. Chaque superpuissance tente d'asseoir son « messinat »- cette alliance du messie et du mécénat. Diplomatie transactionnelle ou intéressée, chacun appréciera. Il n'en demeure pas moins que la France doit pouvoir répondre présente dans les grands défis qui attendent notre monde. Prenons un exemple concret d'une solidarité qui se veut réellement ambitieuse. Le programme Covax prévoit la livraison de plus de 2 milliards de doses de vaccins, d'ici à la fin de l'année, à destination de l'Afrique. Ce programme constitue à lui seul le meilleur antidote au nationalisme vaccinal. Cette mondialisation-là a du sens on n'a pas tous les jours l'occasion de s'en réjouir. Aristote disait : « Réfléchis avec lenteur, mais exécute rapidement tes décisions ». Monsieur le ministre, je crois que nous avons assez réfléchi : le monde nous regarde, il est temps désormais d'agir.

annoncé par le Président de la République en 2017, ce projet de loi a été plusieurs fois reporté. Même s'il intervient très tard, nous avons de bonnes raisons d'y être attentifs. Premièrement, l'article 15 de la loi de 2014 prévoyait une révision cinq ans après sa promulgation.

On ne saurait imaginer qu'une hausse de 36 % sur cinq ans ne s'accompagne pas d'une véritable politique d'évaluation et de contrôle, alors même que la France et ses citoyens doivent supporter les graves conséquences économiques de la crise sanitaire. Troisièmement, le domaine de l'APD connaît une révolution sur le fond et sur la forme. Aussi, la France, en tant qu'acteur traditionnel, doit s'adapter à un contexte évolutif pour se maintenir dans les premiers rangs des pays pourvoyeurs d'aide publique au développement. Il serait dommageable que ce projet de loi devienne un catalogue de bonnes intentions, une transposition de normes idéologiques inadaptées à la réalité du terrain et aux besoins des bénéficiaires de l'APD française. Cette politique ne saurait être la projection de préoccupations propres à la société française et occidentale sur d'autres populations, dont les besoins sociétaux et les modes d'organisation divergent des nôtres. L'aide publique au développement est autant un vecteur de sécurité globale qu'un outil d'influence internationale et diplomatique. Même s'il s'agit de, c'est un nouvel espace de compétition entre les puissances. Rappelons que l'attractivité de l'APD tient autant à son universalisme qu'a son pragmatisme. J'en arrive aux objectifs de notre politique d'APD. Les rapporteurs, que je remercie de leurs travaux, ont souhaité, à juste titre, les clarifier et les hiérarchiser autour de trois thématiques l'éradication de la pauvreté et l'accès aux services essentiels ; ensuite, la protection des biens publics mondiaux dont celle de la planète ; enfin, la promotion des droits humains et le renforcement de l'État de droit et de la démocratie.

Pallier les difficultés des États et renforcer les structures de gouvernances sont des priorités. Nous avons, ici même, débattu des limites de l'opération Barkhane. L'autre point clé du projet de loi qui mérite notre attention est la trajectoire financière. Monsieur le ministre, nous saluons votre démarche, mais nous regrettons, comme d'autres, que votre horizon s'arrête

s'étend jusqu'à 2030. Nous partageons l'approche de la commission des affaires étrangères, qui ne se contente pas d'une vision quantitative fondée sur le volume de crédits, mais qui prône une approche qualitative reposant sur un rééquilibrage entre dons et prêts et entre multilatéral et bilatéral. Ainsi, fixer un seuil minimum pour les dons à 65 % et un maintien de la part d'aide bilatérale à 70 % nous paraît tout à fait juste. Par ailleurs, cette proposition de ventilation en faveur des dons permettra une meilleure visibilité, une meilleure traçabilité, voire une plus grande sécurisation de l'aide française, me semble-t-il. Les prises de participations de l'AFD au sein de banques étrangères de développement ne sauraient incarner la politique française d'aide au développement. concerne le fonctionnement à venir de l'Agence française de développement, dorénavant autorisée à détenir tout ou partie du capital d'Expertise France, notre groupe souhaite rappeler que, si les objectifs de cette réforme structurelle sont d'achever la création d'une véritable holding de développement et de créer des synergies entre les deux opérateurs, la priorité des priorités reste le renforcement du pilotage stratégique. Dans cette perspective, nous approuvons pleinement l'article 9 mettant en place la commission de contrôle et d'évaluation Nous espérons que le premier axe de travail de la future commission sera d'examiner attentivement le projet immobilier baptisé « Réconciliation », dont le montant avoisine les 836 millions d'euros. il sera primordial de veiller à la préservation de l'identité et des missions d'Expertise France au sein du groupe. Monsieur le ministre, mes chers collègues, notre groupe votera ce projet de loi, afin d'amorcer une réforme de l'APD, laquelle ne doit être qu'une première étape vers une tradition de transparence. C'est un effort important, une générosité qui fait honneur à notre pays, mais qui impose de mettre en place, sans plus attendre, un meilleur contrôle et une plus grande transparence des politiques d'aide au développement. La discussion

à M. Guillaume Gontard. L'objectif de cet amendement est d'inscrire dans le corps de la loi la nécessité d'une mise en cohérence de toutes les politiques publiques avec les objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, afin qu'elles contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable, les ODD. Ce principe de cohérence était un acquis important de la loi du 7 juillet 2014, qui disposait qu'« une cohérence est recherchée entre les objectifs de la politique de développement et de solidarité internationale et ceux des autres politiques publiques susceptibles d'avoir un impact dans le domaine du développement Nous regrettons que la version actuelle de l'article 1 A ne fasse qu'une allusion à ce principe de cohérence, sans spécifier ni le rôle de l'État quant à cette cohérence, ni les politiques ciblées par cette dernière, ni son lien avec les objectifs du développement durable.

cette formulation permet de rappeler que cette cohérence est, à ce jour, un objectif que la France doit atteindre, et non une composante automatique de sa politique d'aide publique, comme l'implique l'actuelle version du texte. Cette nécessité de cohérence doit faire l'objet d'un engagement clair de la France, alors que les manquements de la politique française de développement ont, en 2018, été pointés du doigt par l'OCDE lors de sa revue par les pairs. L'OCDE constatait qu'aucun dispositif ne permet de garantir la cohérence des politiques françaises au service du développement durable. Elle en concluait que « La France doit se doter d'un dispositif de gouvernance pour promouvoir la cohérence de ces politiques. Elle doit s'assurer que ses efforts

Cet objectif est nécessaire pour assurer, à terme, l'autosuffisance de ces États, qui ne demandent que cela. À ce titre, l'alinéa 147 du cadre de partenariat global résume assez bien la situation l'Afrique dispose d'une population en croissante augmentation et jeune et, si les conditions étaient réunies, elle pourrait s'affranchir des dépendances qu'elle subit aujourd'hui. D'un autre côté, dans le cadre de sa stratégie commerciale internationale, la France vise l'objectif de favoriser la signature d'accords conduisant à la création de zones franches. Ces dernières, surtout développées en Asie au début des années 1980, avaient vocation à favoriser l'implantation de multinationales occidentales dans les pays dits « émergents ». Ces dernières y bénéficiaient de conditions avantageuses en matière de fiscalité et de rapatriement des profits, mais aussi d'une main-d'oeuvre nombreuse.

ces implantations n'ont jamais servi à faire monter en compétences et qualifications les travailleurs et travailleuses de ces zones. Elles n'ont servi qu'à ajouter un échelon de division du travail par l'externalisation. Deuxièmement, la multiplication des zones franches a freiné le développement des entreprises locales. En effet, ces dernières ne bénéficient pas des mêmes avantages fiscaux et tarifaires, ce qui conduit à un simple transfert de la production. Troisièmement, ces exemptions de taxes et de douanes, voire de changes, grèvent massivement la fiscalité des pays concernés, donc leur capacité d'investissement interne. Il y a clairement un manque de cohérence dans nos politiques extérieures, qu'il conviendra, un jour, de régler. Les dispositions de cet amendement participent de cette volonté de clarification et d'harmonisation, allant dans le sens du narratif de ce projet de loi,

En l'occurrence, s'agissant de l'amendement n° 184, le texte comprend déjà des références précises au principe de cohérence des politiques publiques, dans l'article 1 A lui-même, ainsi qu'à l'article 2 et, de manière très détaillée, à partir de l'alinéa 30 du rapport annexé. Il ne paraît donc pas nécessaire de modifier ce dispositif

d'intervertir les alinéas 2 et 3 du triptyque des objectifs globaux de la politique de développement solidaire. On partirait du plus général, à savoir l'éradication de la pauvreté dans toutes ses dimensions et la lutte contre les inégalités, la protection des biens publics mondiaux et, enfin, la protection des droits des droits humains. Cela correspond, d'ailleurs, à la définition que donne l'ONU des biens publics mondiaux.

Monsieur le président, parler du développement sans aborder la dimension sociale nous paraît tout de même problématique. Les rapporteurs ont choisi de recentrer le préambule autour des objectifs clés de la politique de développement, mais il reste silencieux sur le respect et la promotion des engagements internationaux de la France en matière de protection sociale, alors que la précédente loi de 2014 consacrée au développement et à la solidarité internationale en faisait mention. Ne pas évoquer ce sujet nous semble marquer un recul important, ne serait-ce qu'en matière de développement durable. L'amendement n° 35, présenté amendement est en partie rédactionnel. Il vise à suivre la définition de l'ONU des biens publics mondiaux et, ainsi, à citer

présent projet de loi s'attelle aussi à rappeler les idéaux humanistes de la France. En ce sens, comme le précise l'exposé des motifs, il promeut, dans le cas de la diplomatie féministe de la France, l'égalité entre les femmes et les hommes et entre les filles et les garçons. Il cite également, parmi les droits humains qu'il convient de préserver, les droits de l'enfant. Nous convenons tous de l'importance de ces enjeux au niveau global et de l'urgence dont ils relèvent dans certains cas. Cependant, le texte omet de parler des droits des personnes LGBTQI+, alors que nous savons les droits de ces personnes ne sont pas toujours respectés, ni même reconnus. Le présent amendement a ainsi pour objet d'inscrire de manière explicite l'engagement de la France dans la lutte en faveur des droits des personnes LGBTQI+ dans le monde. Rappelons-le, le rapport du Global Philanthropy Project révèle que la France consacre un effort financier à la lutte contre les LGBT-phobies dans le monde bien inférieur à celui de ses voisins européens.

contre 264 000 dollars pour la France ... Ce n'est pas beaucoup ! Le plan national d'actions pour l'égalité des droits, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ 2020-2023 prévoit que le ministère de l'Europe et des affaires étrangères amplifie son action en faveur de la protection

de loi texte entend décliner la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales portée par la France. Je rappelle simplement que notre pays est le berceau de l'état civil.

de la politique de développement de la France celui de l'enregistrement des naissances et de la mise en place d'état civil fiable. Il s'agit d'un principe directeur de la politique du développement solidaire.

Cet amendement vise ainsi à faire mention des droits qui ont été reconnus aux peuples autochtones par l'Assemblée générale des Nations unies. Il nous sera opposé, comme ce fut le cas en commission, que les droits humains sont universels et prennent déjà en compte les peuples autochtones. Les droits spécifiques reconnus à ces derniers devant la communauté internationale seraient donc superflus. Comment expliquer alors que ces droits aient été fréquemment et massivement violés par certains des projets que nous finançons directement ? Prenons l'exemple du parc naturel de Kaziranga, en Inde, auquel nous avons consacré 80 millions d'euros depuis 2012 et que la ministre de la transition écologique a visité à la fin versé finance notamment le renforcement de l'équipement des gardes forestiers du parc, qui ont pour instruction de tirer à vue sur tous les intrus. Or ces derniers sont aussi, à leurs yeux, tous les habitants de ces territoires, quels que soient l'ancienneté de leur présence, leur attachement à cet environnement et les moyens nécessaires à leur expulsion ... Résultat, depuis vingt ans, 106 personnes ont été tuées à Kaziranga, dont des enfants. Les autres, ceux qui ont accepté l'expulsion, ont perdu une partie de leur identité et de leur culture, car ces populations ont une proximité et un attachement à leur environnement qui n'est pas comparable au nôtre. Malheureusement, ce cas n'est pas isolé, car 80 % de la biodiversité mondiale se trouvent sur les territoires des peuples autochtones. Les aires naturelles protégées ne peuvent donc tout simplement pas être conçues sans ces populations. Par ailleurs, celles-ci protègent leur environnement mieux que quiconque dès lors qu'on leur en donne les moyens, comme l'a reconnu l'AFD en Amazonie. Comment considérer, face à ce bilan, que la simple mention des droits humains permette d'éviter des désastres humains et culturels ? D'autres donateurs importants, comme le Canada, l'Allemagne ou, plus récemment, les États-Unis, prennent davantage en compte les droits des peuples autochtones dans leur politique d'aide au développement.

Or, s'il est vrai que la santé et l'éducation sont aussi, bien sûr, des biens publics mondiaux, dans la mesure où leur renforcement bénéficie à tous, ce sont avant tout des services de base, qui doivent être dispensés à l'ensemble des populations, même aux plus pauvres, et peut-être surtout à ces derniers, dans les pays en développement. C'est pourquoi il nous paraît préférable de conserver leur mention dans le 1°. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable

contre le travail forcé sont des objectifs premiers de l'aide publique au développement française, bien qu'elles constituent des exigences que l'APD doit également, autant que possible, s'efforcer d'atteindre. L'avis de la commission est défavorable.

1 A. Ces principes « sur l'application de la législation internationale des droits humains en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre » ont été présentés le 26 mars 2007 au Conseil des droits de l'homme, puis le 7 novembre 2007, lors d'un événement en marge de l'Assemblée générale des Nations unies coorganisé par l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay. Cependant, l'article 1 A doit rester un article succinct, qui permet de faire référence à l'ensemble des droits humains. Pour éviter tout, il est préférable de ne pas préciser à l'excès ses dispositions. En outre, les principes de Yogyakarta, élaborés au nom d'une coalition d'ONG, n'ont pas de valeur contraignante en droit international des droits de l'homme. Ils n'ont pas été endossés formellement par les États,

205 tend à préciser que la santé et l'éducation sont des biens publics mondiaux. C'est exact, mais ceux-ci constituent aussi des services essentiels dans les pays en développement, ce qui justifie leur présence dans le 1° du présent article. L'avis de la commission est donc défavorable.

j'ai déjà dit à plusieurs reprises que la France promouvait une approche globale des droits humains qui se fonde sur la Charte des Nations unies et sur les principaux traités et conventions en matière de droits humains qu'elle a ratifiés. Énumérer avant l'article 1 du projet

un avis défavorable

qui permet de rappeler l'indépendance de l'aide publique au développement à l'égard de l'action diplomatique et militaire. Pour reprendre les termes d'une ONG que nous avons rencontrée, si l'APD est l'un des piliers de l'action extérieure de la France,

leur inscription dans la durée et leur nature multidimensionnelle et transnationale exigent une approche globale, s'inscrivant dans un continuum d'actions relevant de la diplomatie, de la sécurité, de l'humanitaire, de la stabilisation et du développement. La notion de continuum est au coeur de la stratégie française Prévention, résilience et paix durable » et fait référence à la simultanéité des interventions de tous les acteurs concernés à toutes les phases des cycles de fragilité et de crise, selon une intensité qui varie en fonction des besoins. Ces actions doivent nécessairement être mises en oeuvre de façon complémentaire, raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable

Gréaume. Cet amendement a été déposé pour résoudre un problème de cohérence. Déclarée grande cause du quinquennat, la lutte pour les droits des femmes et l'égalité entre les sexes a par ailleurs été définie comme axe prioritaire et transversal de l'APD française lors du comité interministériel de la coopération internationale et du développement de 2018, puis en 2019 dans une tribune gouvernementale. On aurait donc pu s'attendre à un projet de loi ambitieux en la matière. Or, si le cadre de partenariat global rappelle cette priorité, la France reste encore largement en dessous des standards internationaux. La commission a une nouvelle fois rehaussé le curseur, pour que 75 % de l'aide publique au développement bilatéral comprennent une dimension féministe. C'est une première avancée, mais celle-ci demeure insuffisante à deux titres. Premièrement, on a du mal à voir d'où pourrait sortir cette cible de 75 %. En 2013, la précédente loi de programmation de l'aide publique au développement avait fixé la cible de Le plan d'action de l'Union européenne sur l'égalité des genres dans l'action extérieure 2021-2025, dit « GAP III », fixe une cible de 85 % des projets d'aides intégrant le genre de façon principale ou significative reprenant les marqueurs 1 et 2 de l'OCDE. D'ailleurs, c'est en partant de ce document que des pays comme la Suède ont déployé une politique diplomatique féministe. Aujourd'hui, le retard français interroge, comme le rappelait le Haut Conseil à l'égalité entre les Deuxièmement, il y a une nouvelle fois urgence. Comme le relève le très bon rapport de la délégation aux droits des femmes du Sénat, celles-ci sont une nouvelle fois les premières à souffrir de la crise sanitaire. Que ce soit en matière d'accès à l'autonomie financière et aux droits fondamentaux, notamment en matière d'éducation et de santé, ou dans la lutte contre les violences, la crise pourrait effacer, en une seule année, les vingt-cinq années de progrès réalisées en matière d'égalité entre les femmes et les hommes à la suite de la conférence mondiale de Pékin. Une nouvelle fois, nous devons profiter du présent projet de loi pour faire passer à la France un cap en matière d'appui aux luttes féministes dans le cadre de l'aide publique au développement. Quel

dont le genre est l'objectif premier. C'est ce que nous faisons, par exemple, le lancement d'un fonds de soutien, qui mobilisera, pendant trois ans, 120 millions d'euros pour financer les activités des mouvements féministes dans le monde. Nous ne sommes pas favorables à cet amendement, même si nous prenons

poursuivons le débat sur le concept du continuum 3D. Cet amendement vise à distinguer les actions de coopération militaire du champ des politiques d'aide au développement solidaire.

suffirait à financer les 5,5 milliards de dollars nécessaires pour aider les personnes les plus vulnérables de la planète. Si l'on ramène ce chiffre à l'échelle de la France, qui a son lot d'OPEX et d'actions de coopération, on peut imaginer l'impact

l'avis de la commission ? Cet amendement tend à préciser que les actions de coopération militaire auxquelles participe la France ne constituent pas des actions entrant dans le champ de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

L'objectif de développement durable, l'ODD 16, nous appelle à apporter collectivement une réponse coordonnée aux défis rencontrés par les bénéficiaires, en améliorant l'articulation et la cohérence des actions de différents acteurs relevant de la défense, de la sécurité, de l'humanitaire, du développement, etc. La distinction entre activités militaires et activité d'appui au développement est clairement établie par les règles de comptabilisation de l'APD établies par l'OCDE, auxquelles nous nous conformons. Le financement de matériels militaires et d'activité militaire n'est pas compatible avec l'APD. Si certaines activités de développement conduites par des acteurs de sécurité, comme la formation à la protection civile, par exemple, sont prises en compte dans l'APD, elles sont soumises à des règles très strictes adoptées dans le cadre de l'OCDE en 2016. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement

Souvent sous-estimée, voire oubliée, cette participation est pourtant un aspect essentiel de l'approche par les droits qui est citée dans le cadre de partenariat global, Cette précision est également fondamentale si l'on considère que, dans les pays prioritaires de la France, les moins de 18 ans représentent souvent la moitié de la population. Il s'agit d'un apprentissage à la citoyenneté et à l'émancipation, qui participe du principe « plutôt choisir que subir

l'approche par les droits, qui vise à rendre les bénéficiaires de la coopération-développement acteurs et actrices de leur propre développement,

L'égalité d'accès des filles et des garçons aux espaces de décision ne va pas de soi. La participation des jeunes, celle des filles et des jeunes femmes, doit faire l'objet de mesures spécifiques La participation des filles dans les espaces politiques et économiques, comme dans tous les espaces, doit être encouragée. Elles ont un rôle clé à jouer dans les dynamiques de transformation sociale, y compris dans les positions de leader. leader. Il convient donc de favoriser dès le plus jeune âge le développement du leadership féminin et l'engagement des jeunes, filles et garçons, au travers d'une éducation au leadership et à la citoyenneté qui permette aux enfants et aux jeunes de développer les connaissances, attitudes et compétences nécessaires

est en cohérence avec les avancées inscrites dans le cadre de partenariat global et avec l'approche fondée sur les droits humains des Nations unies, qui vise à rendre les bénéficiaires de toute politique de développement acteurs et actrices de leur propre

de leurs droits et la prise en compte de leur situation et de leurs parcours sociaux spécifiques. De nombreuses jeunes filles et jeunes femmes, des systèmes d'oppression sexiste et des mariages forcés ou une exclusion des sphères de décision, sont écartées de la vie citoyenne de leur pays ou de leur localité. Nous devons, dans le cadre d'une diplomatie féministe cohérente, encourager la participation de toutes et tous, dès le plus jeune âge.

Marie-Arlette Carlotti. Cet amendement vise à demander la participation des personnes en situation de pauvreté et des plus vulnérables à la politique de développement.

que l'on ne peut que partager, s'agissant en particulier de pays où ces catégories sont malheureusement fortement présentes au sein de la population. La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

C'est un projet ancien, dont le coût avait été chiffré, en 2002, à 100 milliards de francs CFA par le Bureau national d'études techniques et de développement, le BNETD, de Côte d'Ivoire. Mais les gouvernements français successifs se sont fait les relais des grands groupes hexagonaux pour aboutir à un projet

ponctionnent ces pays au lieu de les développer. Nous sommes ici au coeur du problème de la cohérence de nos politiques de développement. Le coût actuel du train urbain d'Abidjan représente cinq fois plus qu'il n'en faut

essentiel pour l'exploitation du nickel et du fer, et qui est évalué à 1 050 milliards de francs CFA, pour ne citer que ces exemples. Quel est l'avis de la commission ? Les auteurs

déjà de s'appuyer sur les entreprises locales, mais elle tâche aussi d'obtenir des réponses aux appels d'offres par des entreprises françaises. Certes, il est souhaitable de faire travailler encore davantage les entreprises locales, mais il ne faudrait pas donner l'impression que la France n'est pas attentive aux besoins des pays récipiendaires

est l'avis du Gouvernement ? L'article 1 A rappelle que la politique de développement de la France « veille à s'aligner sur les stratégies de développement des pays partenaires et à répondre aux besoins des populations », conformément au principe

qu'ils représentent la volonté politique des États membres. La France est très respectueuse de ce principe. L'aide liée reste très modeste : elle représente environ 3 % du total des engagements bilatéraux depuis 2010.

nous sommes très attachés, se pose une question très sensible dans le cadre des actions humanitaires et de développement que nous finançons sur le terrain : le criblage des bénéficiaires finaux des projets. La règle générale, c'est que l'action humanitaire implique la non-discrimination, raison pour laquelle nous considérons que le criblage des bénéficiaires finaux de l'action humanitaire ne doit pas être imposé. À l'inverse, dans le domaine du développement, nos opérateurs, notamment l'AFD, sont soumis à un certain nombre d'obligations relatives, par exemple, à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En conséquence, ils sont tenus de veiller au criblage des bénéficiaires finaux. Le problème est qu'il

doivent être appréciées au cas par cas. Je pense notamment aux transferts de cash, directs ou indirects, dans le cadre de projets axés sur l'employabilité des jeunes ou sur la formation professionnelle. Dans ces cas, il existe des risques de

Mme Nicole Duranton. L'alinéa 7 de l'article 1 A inscrit pleinement l'action humanitaire dans la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales de la France. Cet amendement vise ainsi à pleinement intégrer cette phrase, insérée en commission, dans le sujet du volet d'urgence dont traite ce paragraphe. Lors de la dernière Conférence nationale humanitaire, le Président de la République a réaffirmé l'attachement de la France au principe de non-discrimination dans l'attribution de l'aide, suivant les besoins des populations en situation d'urgence humanitaire. Le droit international humanitaire ne porte aucun jugement sur les motifs des combats et ne fait pas de distinction entre les personnes qu'il protège. Tout le monde doit être traité avec humanité. Quant au sujet du criblage appliqué à l'ensemble de l'aide publique au développement, il est justement traité à l'article 13 du présent projet de loi, dans le cadre d'une demande de rapport. En effet, la réflexion sur la doctrine française est encore en mouvement,

nous émettons un avis défavorable sur l'amendement n° 314. L'amendement n° 36 rectifié tend à supprimer la mention du principe de non-discrimination dans l'article 1 au motif qu'il s'appliquerait non seulement en situation d'urgence humanitaire, comme l'a confirmé le Président de la République lors de la dernière Conférence nationale humanitaire, mais aussi, plus largement,

en vue d'adapter les règles en vigueur. Il est effectivement préférable, tout en réaffirmant le principe de non-discrimination pour les situations d'urgence humanitaire, d'attendre les conclusions de ce rapport pour se prononcer sur une extension supplémentaire de ce principe. Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 36 rectifié.

elles ont un effet dissuasif important sur les entreprises. Or la jurisprudence internationale, si elle a admis des extensions au principe de territorialité des sanctions, a rendu un avis clair contre la pratique américaine, au nom de la souveraineté des États. Le principe de souveraineté permet aux États de promulguer des lois éventuellement extraterritoriales, sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux règles de droit international. seule l'extraterritorialité d'édiction est autorisée, mais pas son exécution. Si les États-Unis sont logiquement inéligibles à l'APD, il semble essentiel que la France porte une attention particulière aux pays victimes de l'extraterritorialité.

Une nouvelle fois, il s'agit de renforcer la cohérence de l'APD avec le droit international, d'autant que la colonisation par Israël de la vallée du Jourdain prive les Palestiniens de la moitié de leur territoire, dont son coeur économique et agricole.

? L'amendement tend à inscrire des mentions relatives à la défense de la langue française au sein de l'article 1

l'AFD, afin de soutenir l'éducation primaire et secondaire de 27 pays francophones. Nous avons demandé à l'AFD de promouvoir davantage la francophonie, à l'occasion de l'extension de son mandat aux industries culturelles et créatives, avec un ciblage sur les pays francophones.

Paradoxalement, les personnes en situation de handicap, qui souffrent souvent d'exclusion sociale dans leur pays, sont les grandes oubliées de ce projet de loi. Elles devraient pourtant être prioritaires et bénéficier de notre pleine solidarité.

de handicap sont confrontés à de nombreux obstacles. Ils ne bénéficient pas d'un accompagnement personnalisé, dans le cadre de leur formation et de la réalisation de leur projet professionnel, lorsqu'ils y ont accès.

Cet amendement vise donc à faire en sorte que l'aide bilatérale de la France, qui combat toute forme de discrimination, oeuvre aussi en faveur du respect des droits de l'homme, particulièrement au bénéfice des personnes souffrant de handicap.

Je comprends le souhait de placer l'intégration des personnes handicapées au coeur de l'action de la France pour l'accompagnement des pays en développement dans la construction de sociétés durables et inclusives.

l'un des moyens pour lutter contre la pandémie. Nous savons qu'il ne sera pas suffisant, contrairement aux leçons que l'on est venu nous faire ici. Nous savons aussi qu'il faudra produire des vaccins partout

existe plusieurs blocages concernant la fabrication des vaccins. Premièrement, il y a ceux qui ne veulent pas donner. La France est au rendez-vous du don.

mais, nous, nous n'avons pas attendu l'élection de Joe Biden pour changer d'avis sur la levée des brevets des vaccins contre le covid. Nous faisons partie des organisations qui ont lancé une campagne européenne sur cette question voilà plus d'un an. Vous avez déclaré

C'est d'autant plus regrettable que ce projet de loi, qui nous est annoncé depuis deux ans, est censé traduire en actions concrètes un effort financier considérable en faveur de l'aide publique au développement portée par la France. Nous nous attendions à des perspectives, mais les alinéas consacrés aux objectifs financiers relèvent plus du bilan. L'article 1 constitue le noeud gordien de ce projet de loi de programmation, après l'article 1 A, qui définit en quelque sorte la philosophie de l'aide publique au développement.

monsieur le ministre. Peut-être l'aile progressiste de la majorité présidentielle n'a-t-elle pas eu, une fois de plus, le poids suffisant pour faire fléchir Bercy, dont chacun connaît l'orthodoxie budgétaire,

si vous ne prenez aucun engagement de programmation, c'est que votre objectif d'atteindre le taux de 0,7 % manque de sincérité et n'est qu'un effet d'affichage. Si vous voulez être complètement transparent sur vos engagements, alors vous devez faire vôtre le tableau

qui représentent plus de la moitié de l'aide mondiale au développement, soit des milliards de dollars,

créée en 2010. Dans la foulée, et à l'occasion de la condamnation en cette même année 2017 du fils du président de la Guinée équatoriale et de la confiscation de ses biens en France, à hauteur de 100 millions d'euros, s'est posé le problème de la restitution de ce type d'avoirs, issus de la corruption transnationale. La proposition de loi de notre collègue Sueur, dont j'ai été le rapporteur, a alors pris tout son sens. Elle avait pour but de garantir l'affectation des avoirs illicites confisqués aux pays et aux populations qui en avaient été privés, mais elle est restée pendante à l'Assemblée nationale.

La proposition de notre rapporteur pour avis Jean-Claude Requier de confier les modalités de restitution au ministère des affaires étrangères, par le biais de l'aide publique au développement, mais sur des lignes budgétaires dédiées, au cas par cas et localement, sur des projets clairement identifiés et, pourrait-on dire, labellisés, constitue un premier pas. Il faudra que tout ceci soit clairement identifié et articulé, notamment dans les prochaines lois de finances, car il faut bien avouer que nous marchons- pardon, que nous avançons -lentement sur ce dossier. Certes, les cas ne sont pas si nombreux, mais ils sont très emblématiques, et il est de notre devoir de veiller à respecter les populations spoliées, ainsi que notre engagement d'une restitution responsable.

Ce discours fort et ambitieux a été largement salué et a bénéficié d'une grande résonnance, mais la France est-elle à la hauteur de ses aspirations ? Je ne le pense pas, et l'absence de la dimension sportive dans ce texte le prouve encore une fois. La France doit affirmer une diplomatie sportive durable et pleinement engagée pour le développement solidaire et la lutte contre les inégalités, face à la puissance de nouveaux acteurs sur la scène internationale et en réponse aux diplomaties sportives agressives, à l'image de celle de la Chine et des pays du Golfe, qui financent la construction de stades dans les pays en développement ou le sport professionnel au travers du rachat de clubs. S'il est hors de question de rivaliser avec ces pays,

Notre pays pourrait être leader sur le continent africain, mais aussi en Inde et dans d'autres pays, pour promouvoir une approche pertinente fondée sur le sport sur des sujets aussi importants que la santé, l'environnement, la formation, la gouvernance, l'organisation de grands événements,

Les acteurs sont prêts, les moyens sont présents : pour que le sport devienne réellement l'un des ciments de notre avenir commun, nous devons désormais inscrire explicitement le sport dans ce projet de loi et reconnaître ainsi pleinement le rôle qu'il joue. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la France est belle et grande quand elle est solidaire et généreuse.

Un ventre creux et une tête vide sont toujours une cible privilégiée pour les mouvements terroristes. À cet égard, aucune politique

à des taux très faibles, voire négatifs. Les pays qui bénéficient de cet argent n'utilisent pas leurs quotas de DTS. Des centaines de milliards de DTS dorment ainsi dans les coffres du Fonds

comme horizon définitif pour atteindre la part de 0,7 % du RNB consacrée à l'aide publique au développement. Cet engagement solennel a été pris par la France à la tribune des Nations unies voilà plus d'un demi-siècle, le 24 octobre

Comment applaudir une telle déclaration si nous manquons toutes les occasions de prendre de réels engagements ? Nous ne comprenons pas bien ce qui empêche d'inscrire dans le marbre de la loi un engagement plus ferme, d'autant que cette loi est avant tout déclarative et ne lie pas les mains du futur gouvernement et du futur Parlement. Au demeurant, avec la crise économique qui s'annonce et la probable contraction de notre RNB, cet objectif relatif sera plus facile à atteindre. Pour toutes ces raisons, nous invitons le Sénat à inscrire un objectif plus ferme à l'horizon 2025, afin de consacrer l'ambition du projet de loi. C'est une occasion unique de poursuivre nos efforts et de revaloriser ce pilier essentiel de notre politique étrangère. La

Il est essentiel de conserver l'ambition de 0,7 % du RNB. Ce projet de loi offre une occasion unique de poursuivre la dynamique enclenchée. Investir aujourd'hui dans l'aide au développement, c'est s'assurer que celle-ci constitue réellement un outil d'influence et de puissance, alors que le préambule du cadre de partenariat global (CPG) souligne sa complémentarité avec l'action diplomatique et militaire, ainsi que sa contribution à la politique étrangère de la France. Par conséquent, c'est s'assurer qu'elle dispose des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs, mais aussi pour s'adapter aux défis mondiaux actuels. L'amendement n° 105, présenté

les pays récipiendaires paient aujourd'hui un lourd tribut du fait du manque d'engagement des États. Sur la dernière décennie, ce sont plus de 60 milliards d'euros qui n'ont pas atteint leur cible. Cela représente dix ans de budgets consacrés à l'éducation ou à la santé Au regard des conséquences à long terme de la crise sanitaire que nous pouvons anticiper, les pays en développement ne peuvent plus se permettre d'attendre. Oui, il est heureux que le cadre de partenariat global réaffirme avec force l'objectif d'atteindre rapidement le seuil onusien,

[du] revenu national brut en 2025 », adoptée par l'Assemblée nationale, est directement issue de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies de 1970. Une telle inscription dans la loi répond à une demande forte de la société civile,

Rappelons-le, la plupart des augmentations de l'APD observées depuis 2017 résultent de la comptabilisation de flux qui ne quittent en réalité jamais le territoire français ou, du moins, qui ne représentent pas d'argent additionnel pour les pays en développement. Selon l'OCDE, l'augmentation de 4,2 % de nos apports d'APD entre 2018 et 2019 résultait de l'augmentation des dons en lien avec une hausse du coût d'accueil des réfugiés et du soutien destiné à des instruments du secteur privé. Ainsi, en 2018, près de 16 % de notre aide ne quittait pas le territoire français. Elle était dépensée sous la forme de frais d'accueil de réfugiés, de bourses et de frais d'écolage ou d'allégement de dette. Ces dépenses sont essentielles, mais elles ne relèvent pas de l'aide publique au développement. L'accueil des réfugiés est une obligation de la France au regard du droit international, pas une dépense facultative visant à soutenir le développement des pays bénéficiaires. Les bourses et les frais d'écolage versés pour l'accueil d'étudiants étrangers en France ne contribuent pas au développement des systèmes éducatifs des pays des bénéficiaires de notre aide. Pourtant, ils constituent l'essentiel de notre aide bilatérale à l'éducation. L'éducation de base, qui est pourtant absolument indispensable pour le développement des pays les moins avancés, est quasiment invisible : elle représente 3 % de notre APD totale. On observe aussi une comptabilisation croissante des financements destinés à soutenir des projets du secteur privé.

consacrer 1 milliard d'euros supplémentaires chaque année aux crédits de la mission « Aide publique au développement » permettrait de compenser la comptabilisation de ces flux, qui vont gonfler les chiffres de notre aide sans se traduire par une réelle contribution au développement des pays bénéficiaires. Ce milliard d'euros permet de s'assurer que l'augmentation de l'APD française ne repose pas sur une augmentation des dépenses domestiques.

dons. Entrons dans le détail. Le remboursement des échéances implique une écriture en APD négative équivalente au remboursement du capital et une écriture en APD positive lors du versement du don, qui comprend le capital et les intérêts. Le solde positif pour le calcul de l'APD française équivaut donc au seul montant des intérêts payés par le pays débiteur. En revanche, les refinancements par dons ont un effet significatif sur les composantes de l'APD, puisqu'ils en réduisent la composante par prêts en écriture négative du montant du capital remboursé, tout en augmentant sa composante par dons par l'écriture positive précédemment évoquée. Je le disais, c'est un peu technique ... Ce jeu d'écriture

le volume des dons comptabilisés en APD française tous bénéficiaires confondus, tandis qu'ils réduisent de 10 % en moyenne le volume des prêts nets de cette même APD. Les contrats de désendettement et

ont été lancés lors du G7 de Cologne en 1999 pour annuler, au titre de l'aide publique au développement, la totalité des dettes contractées par les pays pauvres très endettés, les PPTE.

mais il nous paraît important de fixer des cibles à la fois atteignables et compatibles avec les autres objectifs de notre politique de développement, en particulier l'investissement dans les biens publics mondiaux.

étant donné que cet instrument a vocation à toucher les pays les plus vulnérables et à financer les secteurs prioritaires comme l'éducation, la santé ou l'adaptation au changement climatique. Certains pays comme le Danemark ou l'Australie ont une APD exclusivement constituée de dons. La France, quant à elle, fait partie des plus gros prêteurs, dépassée seulement par le Japon et la Corée du Sud. Selon l'OCDE, en 2018, près de 50 % de l'APD brute bilatérale française était versée sous forme de prêts, contre 16 % en moyenne pour l'ensemble des pays du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE. Les recommandations du CAD sont critiques envers cette répartition très inégalitaire. En effet, privilégier les prêts revient non seulement à favoriser comme partenaires de l'APD des pays à revenus intermédiaires, qui ont moins besoin de notre aide, mais également à accentuer la dette de nos pays partenaires. dette de nos pays partenaires. Cette répartition de notre APD n'est pas tenable si nous souhaitons réellement atteindre les objectifs que nous nous fixons avec ce texte. Par conséquent, la réduction des prêts dans l'aide française doit être une priorité afin de lutter contre les inégalités mondiales.

soit 7 810 milliards de dollars. Dans les 76 pays les plus pauvres du globe, la dette a ainsi doublé en dix ans, avec certains cas extrêmes comme l'Éthiopie, qui connaît une augmentation

Cet endettement alimente une course au surendettement, puisque cela freine les pays emprunteurs dans leur recherche d'investissements nationaux massifs et de développement des services publics locaux.

à hauteur de 500 milliards de dollars annuels d'ici à 2030 pour atteindre la cible de l'agenda de l'ONU. C'est d'autant plus important que, trop souvent, on réduit l'aide publique au développement aux PMA à des annulations de dettes. Bien évidemment, ces mesures peuvent être essentielles pour donner des marges de manoeuvre : elles répondent souvent à une situation devenue intenable.

Todeschini. Cet amendement vise à renforcer la concentration des moyens de la composante bilatérale de l'aide au développement française en direction des pays les moins avancés et de conforter ainsi la stratégie française.

Ce serait l'occasion de faire reculer la misère dans cette région et, par là même, de faire reculer le terrorisme qui se nourrit de cette situation. Marie-Arlette Carlotti l'a souligné : nous connaissons les racines du mal et les raisons qui poussent les populations dans les bras des terroristes. C'est la colère des peuples, qui s'élèvent contre la mal-gouvernance et la corruption. Hélas, cette colère se reporte aujourd'hui contre nos forces armées. Aux côtés de notre force Barkhane, l'autre volet de la lutte contre le terrorisme, c'est bien une politique de développement volontariste au Sahel.

Ce chiffre doit nous permettre de traduire l'effort auquel nous nous engageons de concentrer l'aide bilatérale et les dons aux pays les moins avancés, en particulier les pays prioritaires. L'éradication de la pauvreté dans toutes ses dimensions, dont nous faisons notre priorité, n'est pas un objectif crédible s'il n'est pas accompagné d'un ciblage effectif vers les pays et les populations qui en ont le plus besoin. Or notre aide française ne priorise toujours pas les pays les moins avancés, qui concentrent pourtant les poches d'extrême pauvreté dans le monde. Les 19 pays qui ont été identifiés comme prioritaires

L'objectif fixé par la commission de consacrer 30 % de notre aide pays programmable aux pays prioritaires est louable, mais il n'est pas à la hauteur des ambitions de ce texte. Cela représenterait moins de 2 milliards d'euros distribués entre 19 pays. Cette somme fait pâle figure, alors que le FMI déclarait que 500 milliards de dollars supplémentaires devraient être alloués chaque année aux pays prioritaires afin de respecter les engagements de l'Agenda 2030. L'adoption de cet amendement, qui vise à porter cette part à 40 %, traduirait mieux notre volonté de renforcer le ciblage géographique de l'aide et de prendre ainsi les mesures nécessaires à l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes. Vous l'imaginez, mes chers collègues, nous souhaiterions un objectif encore plus ambitieux, mais, dans l'esprit de compromis qui préside à nos débats, nous vous proposons de rehausser ce volume dans des proportions raisonnables, qui restent en phase avec les annonces de M. le ministre. Quel

Avant même la crise sanitaire, des instances onusiennes alertaient sur la stagnation des progrès réalisés ces dernières décennies en matière d'accès à certains services essentiels. La situation de l'éducation était ainsi préoccupante,

Une nouvelle fois, les pays occidentaux ont fait le choix de sacrifier les populations fragilisées. Se pose dès lors la question de la crédibilité du discours de la France en matière d'aide publique au développement. si Paris consacre près de 1 milliard d'euros d'aide bilatérale à l'éducation, en plus de ses contributions aux instances multilatérales, il alloue moins de 2 % de cette somme à l'éducation de base. En parallèle, la France n'a consacré que 2,3 millions de dollars au Fonds d'urgence, devant

Je vous laisse

pour construire les conditions d'un développement durable des États et leur permettre de réduire la pauvreté, d'assurer des services publics et de renforcer leurs capacités. Si les recettes fiscales représentent en moyenne 34 % du PIB dans les pays de l'OCDE, elles sont deux fois moins importantes dans les pays en développement. Au-delà du volume de recettes fiscales récoltées se pose la question de la nature de la ponction fiscale, qui, pour être efficace, gagne à être guidée par des critères de justice sociale n'aggravant pas la situation des populations les plus pauvres et les plus laborieuses, en mettant à contribution les profits du capital local et du capital étranger. Se pose enfin la question de la redistribution des recettes, pour promouvoir une croissance efficace répondant aux objectifs. L'organisation économique internationale en vigueur, qui se traduit par les actuels traités de libre-échange, est un obstacle à cet objectif, puisqu'elle alimente une course au moins-disant fiscal particulièrement avancée dans les pays en développement, à travers des législations

Pour rappel, lors de la quatrième édition du qui a eu lieu au mois de janvier 2021, la France s'est engagée à accroître la part des financements de l'AFD favorables à la biodiversité, en portant à 30 %, d'ici à 2025, la part de la finance climat directement favorable à la biodiversité

Cela nous semble particulièrement pertinent dans la mesure où l'article 1 A consacre la protection des biens publics mondiaux, dont la protection de la planète est la composante principale, comme l'un des objectifs premiers de notre politique d'aide publique au développement.

est à M. André Guiol. Depuis plusieurs années, l'aide mondiale au développement a pris un tournant, en intégrant la problématique du développement durable dans ses stratégies. C'est en particulier le cas depuis 2015, 2015, année où le programme d'action d'Addis-Abeba a insisté sur l'importance des actions en faveur du climat. Les objectifs de développement durable adoptés dans le cadre de l'Agenda 2030 ont confirmé cette orientation. Je n'oublie pas l'accord de Paris, dont l'article 9 promeut la nécessité d'aider les pays en développement à mettre en oeuvre des mesures d'atténuation du changement climatique. La France, en première ligne pour encourager cette évolution, rappelle régulièrement ses engagements. de janvier dernier, lors du, le Président de la République a décidé de porter à 1 milliard d'euros d'ici à 2025 le montant annuel des financements engagés par l'AFD en faveur de la gestion durable de la biodiversité. Dans le cadre du sommet Ambition Climat qui s'est déroulé au mois de décembre 2020, la France s'est également engagée à maintenir le montant de la finance climat

Depuis 2019, la France prône publiquement une « diplomatie féministe » dans les différents forums internationaux, mais celle-ci peine à se traduire de manière concrète dans une véritable aide publique au développement féministe.

Le Canada, la Suède, l'Irlande, l'Islande, pour ne citer que ces pays, dépassent les 80 % d'APD « genre », quand la France peine à atteindre les 40 % en 2017.

de rehausser la part d'APD « genre » pour atteindre 85 %, d'ici à 2025, ainsi que cela est recommandé par les institutions européennes et le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour cela, nous proposons une trajectoire cohérente et graduelle, portant la part d'APD « genre » à 60

Selon une étude du Forum économique mondial de Davos, la covid-19 a fait perdre trente-six ans à la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes.

N'dongo Samba Sylla et la journaliste Fanny Pigeaud, malgré la suppression apparente du compte d'opérations, le Trésor français a maintenu son rôle putatif de garant de la convertibilité du franc CFA à taux fixe,

on peut dire que le compte d'opérations a disparu pour réapparaître sous une autre forme ! Surtout, et c'est là le tour de force du Trésor, cette nouvelle forme est moins onéreuse pour l'État français, car il n'est plus tenu de verser à la BCEAO des intérêts sur ses réserves au taux nominal de 0,75 %, alors que ce nouveau système assure à la France le même contrôle politique

Cette garantie constitue un facteur de stabilité pour le cadre macroéconomique de la zone ; elle est très utile pour la conduite des politiques économiques. Les moindres recettes pour la BCEAO sont susceptibles d'être compensées,

est à M. André Guiol. L'article 1, qui définit notamment les grands axes de la programmation financière de la politique solidaire, précise que les moyens transitant par la société civile devront doubler en 2022 par rapport à 2017.

est une bonne chose : 460 millions d'euros en 2019 contre 241 millions en 2016. Cette évolution positive souligne l'importance du soutien qu'apporte la société civile au développement solidaire l'article 2 introduit en commission le rappelle fort justement. Cet amendement tend à conforter la rédaction de l'article, en précisant que ces moyens devront atteindre « au moins » 1 milliard d'euros. Il est également proposé de supprimer la référence à l'objectif de la moyenne des pays de l'OCDE. Si la France est actuellement en retard au regard de l'effort fourni par les bailleurs issus de ces pays, le contexte de récession économique mondiale pourrait fragiliser la référence à cette moyenne. En effet, compte tenu de la dégradation de leurs finances publiques, les principaux pays de l'OCDE réduisent leur budget consacré à l'aide au développement. C'est le cas du Royaume-Uni qui a choisi de faire passer son budget consacré à l'aide publique

pour atteindre la moyenne des pays du CAD de l'OCDE. La rédaction actuelle est très peu ambitieuse et permet encore une fois, comme c'était le cas pour l'objectif de 0,7 % du RNB, d'afficher un objectif louable, sans prendre d'engagement contraignant.

Reconnaître leur rôle et leur plus-value, comme c'est le cas à l'alinéa 13 de cet article, est un premier pas dans la construction d'une politique d'aide véritablement partenariale, mais il faut désormais dépasser les déclarations de bonne volonté et s'engager à consacrer les moyens qui permettront de bâtir cette politique.

Tous constatent que la France est largement en retard sur la moyenne des pays du CAD de l'OCDE : 4 % de son aide sont dirigés vers et acheminés par les ONG, contre 15 % pour les pays du CAD. La reformulation de l'alinéa 12 vise à donner aux organisations de la société civile les moyens pour que les objectifs de la politique de développement et de lutte contre les inégalités mondiales puissent être atteints dans un cadre véritablement partenarial.

sujet. La commission a accordé une suite favorable à notre amendement qui porte à 1 milliard d'euros la part d'aide transitant par les ONG. C'est une bonne chose, mais nous souhaitons compléter cet engagement par une date cible qui serait 2025.